réserves d'usage. Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, c'est avec émotion que nous avons appris le décès, mardi, de notre ancien collègue Charles Revet, qui fut sénateur de la Seine-Maritime de 1995 à 2019.

Charles Revet fut un acteur majeur de la vie démocratique de son département. Il consacra son énergie, notamment, au rétablissement de la liaison transmanche Dieppe-Newhaven. Élu plusieurs fois député de la Seine-Maritime, cet homme de foi et de conviction devint sénateur en 1995. Membre du groupe des Républicains indépendants, puis du groupe UMP et du groupe Les Républicains,

la commission des affaires économiques et la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, dont il fut vice-président, par sa connaissance des dossiers agricoles, maritimes et d'aménagement du territoire. Son sens politique conjugué à son sens de l'humour et à sa gentillesse a marqué tous ceux qui ont eu la chance, et j'en étais, de travailler à ses côtés. En juin 2013, président du groupe de spiritualité du Sénat et président du groupe France-Saint-Siège, il avait emmené une cinquantaine de nos collègues, de toutes convictions religieuses, au Vatican. Il était resté très marqué par sa rencontre avec le pape François, désigné quelques mois plus tôt. En 2018, il avait écrit un livre intitulé. Le « et pourtant » » était pour lui essentiel. Au-delà de son inquiétude pour notre pays, il évoquait, comme dans la parabole, « ses talents » pour se redresser. C'était l'une de ses dernières contributions à une Nation qu'il a servie pendant plus de cinquante Au nom du Sénat, je souhaite exprimer notre sympathie et notre profonde compassion à sa famille, à ses proches, au président et aux membres du groupe Les Républicains auquel il a appartenu, ainsi qu'à ses collègues et anciens collègues

je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Chacun sera attentif à observer, au cours de nos échanges, le respect des uns et des autres et celui du temps de parole.

Après le temps légitime de l'émotion et du recueillement vient désormais celui des actes, afin de ne plus laisser « la Manche devenir un cimetière », comme l'a déclaré le Président de la République. Au-delà des circonstances de ce drame, c'est bien toute la gestion de notre politique migratoire qui pose aujourd'hui question, en particulier en lien avec notre voisin britannique depuis le Brexit, avec, en toile de fond, le sort en suspens de populations très fragiles, qui restent irrésistiblement attirées par le rêve d'une vie meilleure outre-Manche ou chez nous. Il y a donc urgence. Oui, les réseaux mafieux de passeurs ont une responsabilité dans la multiplication des tentatives de traversée. Mais le verrouillage de la frontière autour de Calais depuis l'accord du Touquet en est aussi une cause structurelle. Les migrants ne doivent pas devenir les victimes de nos arbitrages politiques. Pour notre part, nous pensons que la solution doit d'abord être gérée par la solidarité européenne. Mais elle ne peut s'extraire d'une réflexion plus large sur notre politique migratoire, au regard des tendances de long terme de notre démographie. Comment parler aujourd'hui de façon crédible de réindustrialisation si la main-d'oeuvre venait à manquer ? Comment garantir la pérennité de notre modèle social si notre économie ne peut plus le financer ? le Panthéon accueillait une migrante, Joséphine Baker, qui a su rendre à la France ce qu'elle lui avait donné et plus encore. Monsieur le ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour garantir une politique migratoire plus juste et plus humaine ?

et, bien sûr, notre colère face au drame qui s'est déroulé au large de Calais le 24 novembre dernier. Beaucoup de vos collègues vont poser des questions sur cette crise migratoire, et je leur répondrai bien évidemment. Mais puisque vous avez prononcé ce mot d'introduction, je tenais à m'associer à vos propos.

Nous devons pouvoir accueillir sur notre sol les personnes qui y viennent pour diverses raisons, ce que notre droit reconnaît depuis des temps très anciens, au moins depuis que la République française est une démocratie.

jugeons que le comportement ou les valeurs ne sont pas compatibles avec la République. C'est un travail très difficile, et je peux vous assurer que, loin des pulsions et des réflexes, le Gouvernement est dans la réflexion et dans l'action.

cela a été dit, vingt-sept personnes sont mortes en mer au large de Calais. Vingt-sept personnes : des enfants, des hommes, des femmes, comme Maryam Nuri Mohamed Amin, jeune kurde irakienne de 24 ans, qui tentait de rejoindre son fiancé au Royaume-Uni. Vingt-sept personnes sont mortes : il est de notre devoir collectif qu'un tel drame ne se produise plus. De quoi sont-elles mortes ? D'un étau mortel : d'un côté, la militarisation grandissante de nos frontières ; de l'autre, l'avidité des passeurs qui en profitent. Monsieur le ministre, vous pouvez ériger autant de murs, de barbelés, déployer autant d'avions et de moyens de surveillance que vous le désirez, la détresse, le chaos climatique ou l'oppression continueront de faire se déplacer des hommes et des femmes vers un avenir meilleur. Votre politique fait la fortune des groupes de passeurs. Plus haut sera le mur, plus chère sera l'échelle qu'ils vendront. Ce naufrage doit être considéré comme le drame de trop. Il nous fait honte, comme nous fait honte, parfois, votre politique quotidienne à l'égard des exilés. Les images des tentes lacérées par des forces de l'ordre ou leurs prestataires nous rappellent quotidiennement la réalité de l'attitude de ce gouvernement vis-à-vis des migrants. Votre réponse à ce drame est désormais de déployer Frontex dans la Manche. Après avoir investi des centaines de millions d'euros en Méditerranée pour empêcher les exilés d'entrer en Europe, vous souhaitez déployer des forces pour les empêcher de sortir d'Europe ! Monsieur le ministre, quand allez-vous mettre fin à cette surenchère militaire, aux actes de maltraitance, et enfin travailler à une politique d'accueil digne ainsi qu'à la création de voies légales et sûres de passage ? La parole est à M. le ministre de l'intérieur.

notamment à mettre en place des routes sûres pour l'immigration légale ; enfin, vingt-huit, c'est le nombre de jours de grève de la faim suivis par un prêtre pour dénoncer votre politique. En réalité, vous menez une politique irresponsable, inhumaine et criminelle La parole est à M. Alain Marc, pour le groupe Les Indépendants - République et Territoires. de l'industrie, la SAM, entreprise du bassin de Decazeville à Viviez, fabrique des moteurs pour Renault. Or le tribunal de commerce de Toulouse vient de prononcer sa liquidation, jetant ainsi 333 employés au chômage. Ce bassin industriel, qui comptait 38 000 habitants il y a cinquante ans, n'en a plus que 18 000 aujourd'hui. Cette perte d'emplois est considérable pour ce petit bassin économique. Au-delà des drames humains qui seront la conséquence de cette décision, comment comprendre la décision de Renault de permettre la délocalisation d'une entreprise dans un pays étranger, probablement la Roumanie, au moment où tout le monde a conscience qu'il faut réindustrialiser notre pays ? Pouvez-vous, madame la ministre, nous indiquer ce que compte faire le Gouvernement dans les prochaines semaines ?

le choc est terrible ; vous avez l'impression que votre monde s'effondre ; vous n'êtes pas responsables de la situation ; ni la qualité de votre travail ni votre engagement ne sont en cause, et vous nous trouverez- vous me trouverez -toujours à vos côtés. Depuis maintenant deux ans, avec Bruno Le Maire, avec Carole Delga, présidente de la région Occitanie, avec Arnaud Viala, président du département de l'Aveyron, ainsi qu'avec les parlementaires et les élus du territoire, nous avons cherché un repreneur. Depuis deux ans, l'État a mobilisé tous les outils pour éviter la liquidation judiciaire de l'entreprise et rendre possible cette recherche de repreneur. Notre responsabilité collective est maintenant de donner un avenir aux salariés et au site de Decazeville. C'est ce que nous faisons en demandant à Renault de proposer un accompagnement financier et social exemplaire.

C'est ce que nous faisons, par ailleurs, en mobilisant le dispositif Choc industriel, visant à implanter de l'emploi industriel sur le territoire de Decazeville. Nous l'avons lancé il y a quelques semaines et nous sommes aujourd'hui en contact avec plusieurs entreprises susceptibles de créer de l'emploi.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, aux Antilles, la situation se dégrade et le lien national se distend. La crise sanitaire a exacerbé des problèmes de fond : coupures d'eau potable, chômage endémique des jeunes, vie chère, baisse démographique, excès d'emplois publics, scandale du chlordécone. La crise en outre-mer est aussi politique et démocratique. La première priorité, c'est le rétablissement de l'ordre public par l'État grâce à un soutien total à nos forces de l'ordre. En effet, ce sont des pharmacies, des bureaux de poste et des cabinets médicaux qui sont pillés. Les autorités locales doivent faire front commun avec l'État pour condamner sans réserve les violences. La seconde priorité, c'est de juguler la pandémie et de permettre l'accès aux soins et aux vaccins. ailleurs, il faut absolument rétablir un dialogue de confiance avec les forces vives des Antilles et trouver des solutions structurelles pour revitaliser durablement les territoires ultramarins, auxquels nous sommes profondément attachés. La somme des diversités des outre-mer fait notre culture nationale et notre fierté. Nous devons refonder les termes d'une relation plus équilibrée et plus partenariale. Cela ne se règle pas par une visite ministérielle express trois semaines après le début de la crise, ou à la veille de l'élection présidentielle. quelle est la stratégie du Gouvernement pour nos outre-mer ? Quelles actions concrètes pour améliorer le quotidien de nos compatriotes ultramarins, qui méritent respect et reconnaissance ?

Nous avons pris des dispositions extrêmement dures- il faut bien l'avouer -, mais courageuses : 1 400 soignants ont été suspendus car ils ne voulaient pas être vaccinés. Il n'y a pas de raison que les métropolitains soit mieux vaccinés,

Monsieur le ministre, votre collègue des outre-mer a parlé d'autonomie à une semaine du référendum sur la Nouvelle-Calédonie, qui fait planer une menace d'indépendance. Cette proposition inattendue est inadaptée et ambiguë. Travaillons plutôt sur la différenciation territoriale, comme le propose le Sénat ! Avec les enjeux considérables qu'ils représentent- stratégie indo-pacifique, économie bleue, richesse de la biodiversité nos outre-mer méritent un débat de fond, dans un contexte apaisé. Construisons avec eux leur avenir dans la République française

a décidé, madame la ministre, de supprimer cette possibilité de recrutement par contrat à compter du 1 janvier prochain. Cette suppression sèche du statut de clinicien hospitalier, alors même que le taux de vacance a doublé, voire triplé, dans certains services à la fin de 2021 met en grand péril la continuité des soins des services hospitaliers, notamment dans les hôpitaux dits périphériques, situés dans des territoires désertés par la médecine libérale et souvent victimes d'une surmortalité et d'une moindre consommation des soins liées à l'isolement. Comment justifiez-vous cette décision, qui, en pleine crise, vient fragiliser encore les services subsistants, privant les hôpitaux publics de professionnels qualifiés ? quelles alternatives proposez-vous pour garantir la continuité des soins dans ces hôpitaux publics confrontés à la menace d'une cinquième vague, et alors que les soignants épuisés croulent sous les heures supplémentaires ?

Par ailleurs, nous réformons l'intérim médical, en deux temps. Des travaux préparatoires sont ouverts depuis un mois : une cartographie de la situation actuelle sera dressée et l'organisation de l'accompagnement dans les Puis, dès que possible en 2022, nous appliquerons la réforme avec un contrôle par le comptable public du respect du plafond réglementaire. que nous apportons s'appuie aussi sur un effort sans précédent pour accroître l'attractivité des métiers et des infrastructures hospitalières, avec près de 30 milliards d'euros du Ségur. Le Gouvernement est donc pleinement au rendez-vous.

Maladies infectieuses émergentes. Les inégalités demeurent criantes à cause de l'égoïsme des grandes puissances : 60 % des personnes sont vaccinées dans les pays riches, contre seulement 3 % dans les pays pauvres. C'est une honte ! Monsieur le secrétaire d'État, allez-vous enfin entendre la demande de l'Inde et de l'Afrique du Sud, soutenue par 100 pays et de très nombreuses ONG, de lever les brevets et les droits de propriété intellectuelle, de partager non seulement les technologies sur les vaccins mais aussi les traitements et les tests anti-covid, afin de permettre à toutes et à tous d'être vaccinés ? Cette demande a été défendue avec force hier lors des rassemblements dans toute l'Europe

je le rappelle, nous sommes le seul pays et le seul continent, par rapport à nos voisins et partenaires britannique ou américain, qui clamaient pourtant la solidarité internationale, à ne pas avoir prévu d'interdiction d'exportation. J'insiste, nous n'y avons jamais eu recours. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est l'Europe aujourd'hui qui a exporté dans le monde le plus de vaccins- un milliard de doses au total -et qui en a donné d'ores et déjà plus de 100 millions, dont 67 millions pour la France- et c'est tout à notre honneur. Nous sommes devenus la pharmacie du monde. C'est l'Europe qui vaccine le monde entier grâce à cette solidarité. Nous sommes le continent- nous devrions le célébrer ensemble, madame la sénatrice -qui en fait le plus, et nous avons débloqué au niveau européen

l'Europe. Je vous rappelle que ceux qui ont parlé de la levée des brevets il y a déjà quelques mois- je pense aux États-Unis en particulier -n'ont jamais fait de proposition en ce sens. Pour notre part, nous sommes concrets : solidarité, livraison de doses, production locale

contre le covid sont uniquement utilisées dans dix pays. Il y a un problème : le dispositif Covax ne marche pas ! Je suis ravie d'entendre que, tout à coup, vous découvrez la licence d'office, car cela fait des mois et des mois que le groupe communiste républicain citoyen et écologiste vous fait cette proposition.

Monsieur le ministre de l'intérieur, la tragédie qui a conduit, il y a une semaine, à la mort par noyade dans la Manche de vingt-sept migrants rappelle cruellement que des milliers de personnes essaient, au péril de leur vie, de traverser ce bras de mer pour rejoindre le Royaume-Uni. Qu'importe si les barrières sont toujours plus nombreuses à Calais, son port et aux abords du tunnel sous la Manche, rien n'entame la détermination des candidats au départ, qui connaissent pourtant les dangers de la traversée sur ces canots pneumatiques de fortune appelés, devenus la marque de fabrique de passeurs faisant commerce de la désespérance humaine. La question migratoire est une question ô combien sensible. Ce drame a légitimement suscité une vive émotion que, tous ici, nous partageons. Je veux avoir en cet instant une pensée pour toutes ces vies brisées. Pour autant, il ne s'agit ni de se convertir aux thèses par trop nauséabondes de l'extrême droite, ni de recourir à certains simplismes démagogiques électoralistes comme ceux qui consisteraient à remettre en cause les accords du Touquet, ni de basculer dans l'angélisme béat. Bien au contraire, il s'agit de montrer que c'est le chemin qui combine humanité, responsabilité et coopération européenne qui est la seule voie de passage. Ce chemin, vous nous l'avez rappelé, monsieur le ministre, c'est celui que notre pays, la France, a décidé d'emprunter. Oui, il faut faire face à cette situation de manière raisonnée, soit tout l'opposé de la réaction du Premier ministre Boris Johnson, inacceptable sur la forme et inique sur le fond. Il s'agit d'abord de lutter plus efficacement contre les réseaux criminels de passeurs, qui profitent des populations migrantes vulnérables, les exposant à des traversées maritimes périlleuses vers le Royaume-Uni. Il s'agit également de renforcer la coopération opérationnelle, non seulement sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord, mais également plus en amont en Europe et dans les pays d'origine et de transit. Enfin, la question fondamentale du partage des demandeurs d'asile entre l'Union européenne- la France en particulier -et le Royaume-Uni doit être mise sur la table. Je pense donc profondément nécessaire la coopération européenne. À ce titre, je salue votre initiative d'avoir réuni très rapidement vos homologues européens. À l'issue de cette rencontre avec vos homologues et de la réunion, lundi, du Conseil de défense et de sécurité nationale, pouvez-vous nous préciser, monsieur le ministre, les engagements pris pour lutter toujours plus contre ce trafic insupportable de migrants et pour éviter que des drames humains ne se reproduisent ? La

des circuits financiers, des nationalités et des législations pour l'achat de bateaux. Nous devons absolument mieux coopérer. C'est ce que nous avons fait dimanche à Calais : pour la première fois, les ministres de l'intérieur se sont réunis sur cette question, qui sera à l'ordre du jour, sur la demande de la France, du Conseil des ministres de l'intérieur et de la justice du 9 décembre prochain à Bruxelles.

la ministre chargée de l'autonomie, je ne peux que rappeler que le contexte de l'actuelle vague épidémique nous donne raison concernant la vaccination obligatoire. Et pour différente que soit la situation dans son pays, le choix du futur chancelier allemand en faveur d'une obligation vaccinale prise sur la base d'une initiative parlementaire, que vous avez pour votre part refusée, ne fait que le confirmer. Dans un autre registre, les informations relatives à la santé des enfants sont aujourd'hui préoccupantes. Elles incitent la Haute Autorité de santé à recommander la vaccination prioritaire des enfants de moins de 12 ans à risque de développer une forme grave ou vivant dans l'entourage de personnes vulnérables. Il y a deux jours en effet, 69 enfants de 0 à 9 ans étaient hospitalisés du fait de la covid-19, et 53 de 10 à 19 ans. Si depuis le début de l'épidémie, il n'y a eu, si j'ose dire, que 13 décès d'enfants de 0 à 19 ans, nous en comptons 9 depuis la mi-juin, et 3 ces dix derniers jours. Nous considérons tous ici que c'est beaucoup trop. Si l'erreur a été commise de confondre moindre risque pour les enfants avec absence de risque, les données qui nous sont présentées aujourd'hui ne nous y autorisent plus. Je rappelle, par ailleurs, que les enfants peuvent également subir les séquelles du covid long et les traumatismes liés à la crainte d'être à l'origine de la contamination des proches vulnérables. Dans ce contexte, le choix de laisser circuler le virus au sein des écoles et de favoriser la continuité en maintenant les classes ouvertes au-delà du raisonnable n'est plus recevable. C'est la raison pour laquelle je vous demande, madame la ministre, quels sont les moyens que vous choisissez de déployer et à quelle échéance pour minimiser le risque à l'école.

dans tous les pays, notamment en Europe de l'Est et du Nord. Notre pays n'est plus épargné par cette cinquième vague épidémique violente, vous le savez, avec un taux d'incidence en hausse forte, désormais supérieur à 300. Le nombre d'admissions pour covid à l'hôpital, y compris en soins critiques, progresse ; la situation reste tendue en outre-mer par ailleurs, un nouveau variant préoccupant, l'omicron, a été identifié. Notre pays prend donc les mesures proportionnées à chacune des étapes de cette crise sanitaire. d'Afrique australe, où le variant fut détecté, sont suspendus jusqu'à samedi. De nouvelles mesures aux frontières ont également été annoncées ce midi par le porte-parole du Gouvernement. Plusieurs cas ont été observés en Europe, dont un cas en France, à La Réunion. Pour contenir son développement,

nous avons ouvert le rappel vaccinal à tous les adultes, à partir de cinq mois après la précédente injection, sur la base de nouvelles recommandations de la Haute Autorité de santé. En pratique, cela concerne 25 millions de Français, dont 7,7 millions ont déjà fait leur rappel. Pour mener cette vaste campagne, il nous faut la mobilisation de tous. Nous comptons sur les médecins libéraux, les pharmaciens, les infirmiers, qui seront valorisés pour cela. Nous réarmons plusieurs centaines de centres de vaccination partout en France. Le rappel vaccinal sera intégré au passe sanitaire. Nous réactivons aussi la ligne prioritaire pour les personnes âgées et fragiles qui ne trouvent pas de rendez-vous immédiat. Bref, le passe

la réplique. Madame la ministre, vous n'avez visiblement pas entendu ma question, à laquelle vous n'avez absolument pas répondu, quelle que soit la mauvaise humeur dont vous faites preuve à l'instant. Je vous parle simplement des écoles, où depuis le début de la crise règne une certaine cacophonie. Croyez-moi, nous gardons beaucoup de modestie parce que nous savons que les choix les choix sont particulièrement difficiles en cette période. Mais il existe aujourd'hui des techniques, notamment des techniques de, qui permettraient de mieux traiter les enfants et de mieux encadrer cette question. La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour le groupe Les Républicains.

à fait ! Je souhaite souligner à quel point cette réponse montre que vous n'avez saisi ni la gravité du sujet ni ses enjeux locaux et nationaux. Vous venez d'indiquer que votre agitation pendant un an n'a conduit à aucun résultat. Ce matin, plusieurs milliers de personnes ont manifesté pour soutenir les salariés de l'usine SAM de Viviez, car « le choc est terrible ». Oui, vous avez raison, le choc est terrible. Vous avez dit que le rôle de l'État est d'accompagner tous les acteurs de la filière- salariés, sous-traitants, constructeurs et équipementiers -, mais nous constatons en Aveyron qu'il n'en est rien. Le cas de la fonderie SAM en est la preuve. L'heure est aux choix, madame la ministre. Choisir l'économie française, c'est vouloir l'implantation en France de productions stratégiques et investir pour leur avenir. Le Gouvernement fait visiblement un autre choix, celui de l'abandon des outils industriels dans nos territoires. Ce choix est incompréhensible et inacceptable pour les 1 000 familles concernées par cet abandon. Ce choix est aussi inquiétant pour la France. Je ne doute pas que les Français ne l'oublieront pas en 2022. Ma question est donc simple, madame la ministre : que dites-vous aux 333 salariés de la SAM pour leur expliquer que la réindustrialisation de la France peut encore attendre ? Que dites-vous aux Français pour expliquer l'incapacité du Gouvernement à sauver le pays ? Et surtout, ne nous dites pas que, pour trouver un travail, les salariés de la SAM n'ont qu'à traverser la France comme on traverse la rue ! L'outil industriel et ses salariés sont en Aveyron, ils doivent rester en Aveyron

a été totale depuis deux ans pour retrouver un repreneur. On aura tout entendu ! Et ce n'est pas la première fois, car nous avons sauvé cette fonderie il y a cinq ans, en 2017. À chaque fois qu'il y a eu des propositions de repreneurs, nous nous sommes mobilisés pour les accompagner et les financer. À chaque fois que des options ont été écartées, nous avons tout mis en oeuvre pour construire des projets alternatifs viables. Vous-même, en mai dernier, avez

question que je pose ! La réindustrialisation, monsieur le sénateur, demande de penser l'industrie de demain, de créer des emplois durables et transmissibles d'une génération à une autre. C'est notre combat au quotidien, avec Bruno Le Maire. Avec France Relance, 24 projets de modernisation pour la fonderie automobile ont déjà pu être soutenus en France, pour 55 millions d'euros d'investissements. De manière globale, 620 projets de relocalisation ont déjà été soutenus partout en France, avec le plan de relance, ce qui va permettre de conforter

Merci de votre réponse, madame la ministre, mais votre parole vous engage. Nous avons trop entendu de promesses non tenues. Je me souviens

C'est à l'État d'intervenir, et nous attendons vos actes ! La parole est à M. Joël Bigot, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous sommes stupéfaits par l'amendement « StocaMine » défendu par le Gouvernement dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances.

adopté sans débat à l'Assemblée par une majorité aphasique, avec comme seule explication du Gouvernement une phrase laconique. Nous relayons ici les inquiétudes des habitants de produits toxiques dans la nappe phréatique d'Alsace, située juste au-dessus du lieu de stockage. L'une des plus importantes réserves d'eau douce souterraine d'Europe est potentiellement menacée par cette décision contraire au principe de précaution. C'est de la santé des générations futures qu'il est question, madame la ministre

Lors du grand débat, le Président de la République avait lui-même reconnu la nécessité d'évacuer le maximum de déchets. Madame la ministre, vos prédécesseurs penchaient à juste titre du côté du déstockage, de préserver la nappe phréatique. Aucun élu ne comprend votre rigidité. N'est-il pas temps de reconsidérer votre position et de reprendre ce dossier en compagnie des élus locaux, afin de rétablir un climat de confiance avec la population et d'éviter ainsi un possible désastre écologique ?

de sécuriser et de donner une garantie financière aux dépenses liées à la sécurisation du stockage. Il s'agit donc non pas de la remise en cause du contexte technique, mais vraiment de la capacité financière de la société des Mines de potasse d'Alsace.

pour une durée illimitée ces produits dangereux en couche géologique profonde. Cela permettra de sécuriser ce site, là où l'affaissement des galeries nous mettait dans une situation très incertaine. Avec cette base législative, nous allons donc pouvoir mener les opérations de mise en sécurité dans les meilleurs délais. La parole Alors que la population vous demande une protection maximale, vous proposez des bouchons de béton dont on n'est pas sûr de la fiabilité à long terme.

Républicains. Monsieur le ministre de l'agriculture, nos agriculteurs sont à bout, et le Conseil d'État vous somme de continuer à les assommer ! Vous avez six mois pour le faire. Vous voulez lutter contre le mal-être des agriculteurs. Pour cela, vous avez annoncé la suppression des termes « mise en demeure » inscrits sur les courriers qui leur sont parfois adressés - car, c'est vrai, cette expression est anxiogène. Et pourtant, le Conseil d'État vous somme encore de les mettre en demeure : mise en demeure d'interdire, ou de limiter au maximum, l'utilisation des produits phytosanitaires sur les sites Natura 2000 Les agriculteurs avaient accepté le zonage Natura 2000 il y a vingt ans, car il partait d'un bon principe : si les pratiques agricoles n'avaient pas d'impact sur leur environnement, elles étaient maintenues. La récente décision du Conseil d'État remet en cause cet équilibre, sans aucune raison ni aucune étude d'impact.

De très nombreux agriculteurs sont donc concernés. La ministre de la transition écologique a même soutenu devant le juge que les activités susceptibles d'avoir une incidence sur les sites Natura 2000 sont soumises à une évaluation, ce qui leur permettait donc d'être conformes à la directive européenne. Or le juge estime, quant à lui, que cette évaluation ne permet pas de s'assurer que l'utilisation des produits phytosanitaires est réduite, voire interdite dans les zones Natura 2000. C'est totalement inadmissible. On assiste, une fois de plus, à une décision dogmatique. On assiste, une fois de plus, à une vraie surtransposition. Quel pays européen s'impose ce jusqu'au-boutisme ? Aucun ! Alors monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour stopper cette énième mise en demeure ?

qui peuvent y être menées sont définies dans les territoires. Vous l'avez dit, le Conseil d'État a pris la décision de nous demander de revoir la mise en application des directives européennes régissant ces zones, eu égard notamment à l'utilisation des produits phytosanitaires.

Ce chiffre descend même à 2035 si l'on retire l'apport de l'immigration. Il s'agit d'un véritable coup de tonnerre, quand on sait que notre pays avait l'un des taux de fécondité les plus élevés d'Europe. Cependant, cela ne nous étonne pas, car nos politiques en faveur de la famille se sont considérablement affaiblies ces dernières années. Après avoir détricoté le principe universaliste des allocations familiales en 2015, les pouvoirs publics ont abandonné les familles dans leur recherche de modes de garde pour nos enfants.

de financement, pour les réinjecter ailleurs, comme on déplace un livre mal rangé dans une bibliothèque. C'est incompréhensible ! Notre modèle se fragilise, et cela dans l'indifférence générale. Monsieur le secrétaire d'État, qu'attend le Gouvernement pour réagir ? Il nous semble urgent de réunir l'ensemble des partenaires sociaux et les associations familiales pour impulser une nouvelle politique familiale ambitieuse pour notre pays. La parole

dans l'ensemble des pays d'Europe, et même au-delà - je pense notamment aux États-Unis. En outre, la France reste le pays au taux de fécondité le plus élevé d'Europe : 1,83 enfant par femme. Enfin, le désir d'enfant dans notre pays reste très élevé, avec près de 3 enfants désirés. Alors, comment expliquer

entre les prestations familiales, le quotient familial et le taux de fécondité. Quel facteur joue sur le taux de fécondité d'un pays ? C'est la capacité d'un pays à créer les conditions d'un accueil favorable

fait d'aider les familles les plus fragiles, avec, par exemple, l'augmentation de 30 % du complément de mode d'accueil pour les femmes seules ou la construction d'un service public des pensions alimentaires et d'un service public de la petite enfance, que nous sommes en train de bâtir pas à pas. Voilà, monsieur le sénateur, le contenu de la politique familiale que nous mettons en place depuis quatre

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, la commissaire européenne à l'égalité, Mme Dalli, a publié un guide interne pour la communication inclusive. Je passe sur le langage non « genré » pour retenir sa dernière initiative : ne plus utiliser le mot « Noël » et les prénoms « chrétiens », qui feraient trop référence à la culture occidentale. Il faudrait les remplacer par des mots neutres et des prénoms reflétant la diversité. Ainsi, « Marie » ne peut plus « partir pour les fêtes de Noël », mais « Rayane » aura le droit de « profiter d'une période de vacances Cette initiative serait risible si elle n'était la partie émergée d'un courant nauséabond travaillant insidieusement à déconstruire la culture européenne au profit d'un leurre transcivilisationnel. Cela va se nicher jusque dans le, qui fait aujourd'hui l'apologie du «

c'est une exhortation que je vous adresse. Allons-nous longtemps continuer à nous laisser dicter notre conduite et notre vocabulaire par la technostructure nocive de Bruxelles, laquelle n'a de cesse de vider de son contenu ce qu'il reste de la civilisation européenne,

Angèle Préville, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Aujourd'hui, à Viviez, à Decazeville et dans tout le bassin industriel alentour, c'est ville morte ! Les commerçants ont baissé le rideau et toute la population- citoyens et élus -retient son souffle, dans une mobilisation sans précédent, appuyée par des dizaines de milliers de citoyens venus de la France entière. ministre chargé de l'industrie, le grand « cri muet » de ce territoire meurtri ? Déjà, en 1987, 3 000 emplois sidérurgistes et métallurgistes avaient disparu. Connaissez-vous vraiment, madame la ministre, ce territoire rural et industriel, qui a perdu des milliers d'habitants en trente ans ? Depuis le 26 novembre dernier, la Société aveyronnaise de métallurgie, la SAM, est en liquidation judiciaire et 333 salariés viennent de perdre leur travail. Le groupe Renault a fait savoir par voie de presse, sans avertir les salariés, qu'il ne soutiendrait pas le projet de reprise. Il est pourtant le seul client C'est donc toujours le même scénario : on s'approvisionne là où la main-d'oeuvre est moins chère, au seul bénéfice des actionnaires :, ce n'est ni plus ni moins que la mise à mort d'un territoire. Les salariés d'abord, mais aussi tous les habitants, vont payer une fois de plus le prix fort. C'est un profond sentiment d'abandon et d'injustice qui étreint ce territoire. La situation de la SAM constitue l'exemple même de la désindustrialisation, organisée par un groupe automobile français, avec la complicité du Gouvernement, principal actionnaire. il s'agit bien d'une capitulation, après deux ans de recherches, en vain, d'un repreneur ! La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, s'est déplacée lundi dernier à Viviez, afin de réaffirmer le soutien de la région à la fonderie, s'engageant d'ores et déjà concrètement pour l'avenir de ce site. De votre côté, vous assistez, résignée, à la fuite inexorable de nos savoir-faire à l'extinction de cette filière d'excellence qu'est la fonderie. Vous affirmez avoir l'industrialisation au coeur, madame la ministre, mais quel est le sens de votre politique ? Combien d'entreprises comme la SAM allez-vous encore abandonner ?

c'est de trouver une solution pour chaque salarié. Cela suppose, d'abord, que Renault prenne toutes ses responsabilités. C'est ce que nous avons demandé, afin que ce groupe propose un accompagnement individuel à chaque salarié.

Enfin, je l'ai indiqué à deux reprises cet après-midi, nous travaillons à l'accélération des projets de développement industriel du territoire, avec le dispositif Choc industriel, que nous avons déclenché. Nous sommes donc en contact avec un certain nombre d'entreprises ; nous avons des projets de créations d'emplois sur le territoire et nous espérons pouvoir ouvrir ces emplois aux salariés de Decazeville. Toutefois, vous le savez, il faut aller plus loin. Ce qui est en jeu, c'est l'accompagnement de la transformation environnementale de la filière automobile. Ce qui est en jeu, puisque vous avez à coeur le combat contre le réchauffement climatique, c'est le fait de passer du moteur thermique au moteur électrique. Ce qui est en jeu, c'est non

La neutralité est donc la règle et le sport s'en trouve pacifié. La Fédération française de football (FFF), par respect pour les valeurs du sport, a également décliné le principe de neutralité dans ses statuts. Ce n'est que la traduction d'une conception du sport qui porte un message universel transcendant les clivages, de quelque nature qu'ils soient. Jusqu'à une période récente, c'était la position de la France

l'interdiction explicite du port de signes religieux ostensibles dans les compétitions organisées par les fédérations sportives, ainsi que l'interdiction de toute forme de propagande religieuse. Ces amendements, adoptés au Sénat malgré l'avis défavorable du Gouvernement, ont été supprimés à l'Assemblée nationale. Les conséquences ne se sont pas fait attendre : des « hijabeuses » ont demandé à la Fédération française de football de revenir sur les principes de neutralité inscrits dans ses statuts. Cette demande a été rejetée par la FFF, et on ne peut que s'en féliciter

En même temps, mon expérience de sportive et de citoyenne française venue d'ailleurs m'impose de défendre le rôle essentiel du sport dans l'apprentissage de la tolérance, de l'acceptation et de la « sublimation » des différences, dans l'appropriation des principes républicains républicains et dans l'émancipation des individus, notamment des femmes. Les enjeux sont plus complexes, en tout cas moins simplistes, que ce que vous décrivez de l'action de l'association qui dépose effectivement un recours devant le Conseil d'État

engageront plus fortement les fédérations aux côtés de l'État, dans un lien plus fort avec les clubs, dans le cadre d'une véritable stratégie d'entrave et de lutte contre le séparatisme.

et des bénévoles. Je compte enfin sur la vigilance des élus dans les territoires, et je suis sûre que, avec tous les nouveaux éléments issus de cette loi, nous saurons lutter efficacement contre le séparatisme dans le sport et ailleurs, ... Il faut conclure ! ... tout en continuant à laisser le sport jouer son rôle émancipateur. Il

pour notre part, nous continuerons de mener un combat sans ambiguïté et sans faiblesse contre l'embrigadement religieux et le repli communautaire, et nous poursuivrons notre lutte sans merci pour l'égalité entre les hommes et les femmes. La parole est à M. Sébastien Meurant, pour le groupe Les Républicains.

les ministres, que ce juge, vice-président d'un syndicat et secrétaire national d'un parti d'opposition, mette en lumière l'échec de votre politique de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, le fond de l'affaire réside précisément là : dans votre refus de vous opposer sérieusement à la fraude. Comme François Hollande naguère, vous semblez considérer que « cela ne coûte rien, c'est l'État qui paie Mais comment expliquez-vous que la France, qui a 67 millions d'habitants, compte 75 millions d'assurés sociaux ? L'argent de la République pousserait-il sur des arbres irrigués par des retraités centenaires vivant au Maghreb ? Dans tout autre pays, un magistrat qui indiquerait au Parlement et au Gouvernement le moyen d'économiser autour de 80 milliards d'euros par an recevrait une promotion et toutes sortes d'honneurs. Chez nous, comme disait Chamfort, « on laisse en repos ceux qui mettent le feu et on persécute ceux qui sonnent le tocsin pourquoi ne vous saisissez-vous pas de ce levier pour améliorer nos comptes sociaux sans mettre à contribution les Français honnêtes et travailleurs ? Y a-t-il une raison cachée à ce refus de s'opposer sérieusement à la fraude sociale ? je sais trop bien que vous refuserez de répondre à la question de fond- nous l'avons déjà posée, ici ou à l'Assemblée nationale, mais en vain, ce qui pose un problème démocratique -, permettez-moi de vous poser une question plus simple et à laquelle on ne peut répondre que par oui ou non : allez-vous mettre un terme à cette procédure scandaleuse contre le magistrat Charles Prats ? La

Monsieur le sénateur, vous interrogez le Gouvernement sur deux points. Le premier relève de la compétence de M. le garde des sceaux, dont je vous prie de bien vouloir excuser l'absence et qui vous aurait indiqué, comme il l'a fait à l'Assemblée nationale, que, à l'heure où nous parlons, le magistrat que vous avez cité fait l'objet d'une enquête administrative qui n'a aucun lien ni avec une activité politique ni avec une décision juridictionnelle. Il s'agit d'une enquête interne visant à permettre au garde des sceaux d'apprécier l'opportunité, sans rien préjuger de la suite, d'ouvrir une procédure disciplinaire pour des faits qui ne relèvent, je le répète, ni de son activité politique ni de son activité médiatique.

la lutte contre la fraude fiscale et permettant d'aller plus loin qu'auparavant, notamment en allégeant ce que l'on appelait, souvent à tort, le « verrou de Bercy ». C'est ce gouvernement qui, en étendant à la fraude fiscale des procédures comme la convention d'intérêt judiciaire

Vous évoquez 8 millions d'assurés indus. Il y a 150 000 cartes surnuméraires, que nous faisons en sorte de repérer, sachant que derrière chaque carte ne se cachent pas forcément des prescriptions. Nous faisons aussi en sorte de lutter contre la fraude à l'immatriculation. Là aussi, les résultats sont au rendez-vous. Les fraudes,

Je rappelle que la discrimination politique est un délit pénal puni par les articles 225-1 et 225-2 du code pénal. Cas unique en Europe, nous avons un ministre de la justice mis en examen. La mansuétude inhabituelle des médias encouragerait-elle le Gouvernement à prendre le risque que celui-ci se retrouve également devant la Cour de justice de la République ?

La séance est reprise. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2022 n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun. L'ordre du jour appelle la désignation de membres d'une mission d'information et d'une commission d'enquête. En application des articles 8 et 8 , alinéa 5, du règlement, les listes des candidats remises par les groupes politiques pour la désignation des membres de la mission d'information sur le thème « La judiciarisation de la vie publique : une chance pour l'État de droit ? Une mise en question de la démocratie représentative ? Quelles conséquences sur la manière de produire des normes et leur hiérarchie ? » et de la commission d'enquête sur le thème « La santé et la situation de l'hôpital en France » ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, incendies, tirs, pillages, violences urbaines, barrages et rackets rythment depuis plus d'une semaine le quotidien des Français en Guadeloupe et, désormais, en Martinique. Ces territoires sont revenus à l'avant-scène médiatique, en raison des menaces et des agressions dont ont fait l'objet les personnels médicaux et non médicaux, ainsi que des entraves à la circulation paralysant l'accès aux soins et mettant en péril la vie de certains patients. Le climat d'insécurité est réel. Professionnels de santé, pompiers, forces de l'ordre, journalistes et photographes sont pris pour cibles par les émeutiers avec des armes lourdes, des pistolets mitrailleurs, des tirs à balles réelles, des coups de feu et des projectiles. Après l'envoi de renforts de police et de gendarmerie- je profite de l'occasion qui m'est donnée pour leur exprimer mon soutien -et l'établissement d'un couvre-feu, la question de l'autonomie vient d'être hâtivement posée sur la table des discussions. En tant que fille d'un Martiniquais habitant au Diamant, je suis choquée autant par la situation actuelle que par la proposition faite. Cette façon d'abandonner potentiellement ce territoire à son sort confirme en effet l'incapacité du Gouvernement à trouver des solutions. Les sénateurs du groupe Union Centriste attendent une politique transversale tenant compte des besoins propres des territoires et des acteurs ultramarins. Mon groupe appelle le Gouvernement à répondre en profondeur aux raisons de la colère des Guadeloupéens et des Martiniquais, dont la crise sanitaire n'a été que le détonateur. Les facteurs sous-jacents à cette crise sont en effet d'ordre social et économique. La contestation vaccinale n'est que la partie visible de l'iceberg. Il semble que le Gouvernement passe à côté de la réponse attendue par la population ultramarine, à savoir une réponse plus économique et sociale que sanitaire. L'obligation vaccinale est la « goutte d'eau qui a fait déborder le vase », même si je n'approuve pas une telle résistance à la vaccination. sanitaire, une série de revendications concernant l'emploi, l'eau, le pouvoir d'achat, le prix des carburants et du gaz, le mal-être social et économique. Accablée par les émeutes de rue, la population attend d'abord le retour au calme. Il est indispensable de rétablir l'ordre public pour permettre à nos îles de reprendre une vie normale et d'engager des discussions. Le blocage des réseaux routiers perturbe l'activité économique, la libre circulation des habitants et la livraison des marchandises, entraînant des phénomènes de pénuries de produits de consommation de première nécessité dans certaines communes. une image catastrophique au regard de la saison touristique. Les touristes n'osent pas sortir de leur chambre d'hôtel et avancent leur date de retour pour éviter le risque d'être de nouveau bloqués sur l'île. Alors que la haute saison approche, l'activité des agences de voyages est complètement à l'arrêt. On note un ralentissement des réservations au départ de l'Hexagone et une augmentation des annulations. Il convient d'élaborer un plan de reconquête du tourisme en outre-mer, pour éviter l'effondrement de l'économie touristique. L'État doit se donner les moyens de sauver l'économie des outre-mer. Face à la situation explosive que connaissent les territoires d'outre-mer, il convient de faire confiance aux élus locaux, pour trouver, collectivement, Il est temps de réfléchir à un plan pluriannuel « Ségur outre-mer » révisant les modes de financement de l'hôpital public, notamment ses moyens humains et ses équipements. Il est temps de poser sur la table un nouveau modèle de développement pour les Antilles françaises, fondé sur la production, ainsi que sur des mesures fiscales. Par ailleurs, d'autres sujets, comme la place de la jeunesse et son avenir dans la société ou les réflexions institutionnelles sur le statut de la Guadeloupe et la gestion économique, ainsi que les perspectives à quinze ans ou vingt ans de ces territoires, doivent faire l'objet d'un dialogue structurant. Ces sujets nécessitent d'être approfondis.

du logement, de la création d'emplois pour les jeunes, de l'encouragement de la production locale et de l'autosuffisance alimentaire et, enfin, de l'adaptation aux fragilités structurelles économiques et sociales. Il ne faut pas prendre ce mouvement social à la légère. Je suis d'ailleurs persuadée que tel n'est pas le cas. En effet, si on remet, une fois de plus,

Madame la présidente, monsieur le ministre- vous arrivez des Antilles -, mes chers collègues, il est difficile d'aborder la question ultramarine sans commencer par dire notre inquiétude quant aux événements qui se déroulent actuellement en Guadeloupe, et plus largement aux Antilles. Il est fait état de barrages, de nuits de violence et de tirs d'armes à feu. Tous les témoignages sont édifiants ! Il faut retrouver le chemin d'un dialogue apaisé, plutôt que de poursuivre une escalade violente. Surtout, le rétablissement de l'ordre public est un impératif que notre groupe soutient sans réserve aux côtés du Gouvernement. Il va également sans dire que les membres de mon groupe, au premier rang desquels Stéphane Artano, qui préside la délégation sénatoriale

On pense forcément au scandale du chlordécone, qui a marqué durablement les esprits. Par ailleurs, nos compatriotes ultramarins sont frappés par des difficultés concrètes souvent inadmissibles et résultant d'investissements depuis trop longtemps insuffisants en matière de services et de politiques publics. Il faut notamment se souvenir que, voilà quelques mois, nous adoptions ici une loi rénovant la gouvernance des services publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe. Ces derniers jours encore, je lisais un article de presse qui redisait combien, sur ce territoire, les habitants sont excédés par les coupures d'eau incessantes. À toutes ces problématiques déjà complexes, une autre question s'est ajoutée, celle du statut de ce département d'outre-mer. Si certains souhaitent une collectivité plus autonome, ce qui aboutirait à revenir sur la position exprimée par la population guadeloupéenne en 2003, une telle revendication n'émane pas de ceux qui se défient aujourd'hui de la politique vaccinale. je comprends l'importance d'un tel sujet ; je comprends que la crise actuelle invite chacun à s'interroger sur le sens à donner au lien entre l'État et cette collectivité. Toutefois, je crois qu'il est prématuré d'aborder le sujet de l'autonomie dans de telles conditions. Cette discussion doit être menée dans un esprit de sérénité, sans violence et dans la concertation, afin de rechercher un équilibre. L'enjeu est trop important pour agir dans la précipitation et ajouter de la tension. Il nous faut sortir de la logique d'urgence et de réaction aux crises. Les territoires ultramarins requièrent un travail de coconstruction des politiques publiques, qui s'effectuerait à long terme et en collaboration avec les acteurs de chacun des territoires. Car, plus largement, les cas guadeloupéen et martiniquais sont symptomatiques des rapports difficiles qu'entretient notre nation avec ses collectivités d'outre-mer. De nombreux efforts devront être fournis. Bien évidemment, les situations sont très variées d'un territoire à l'autre. Cela étant, les outre-mer souffrent, depuis des décennies, de divers déficits en ce qui concerne l'accès aux services publics. Enfin, vous le savez, le Sénat a choisi de mettre à l'honneur ancien président Gaston Monnerville, à l'occasion de la commémoration des trente ans de sa disparition. Aussi, j'achèverai mon intervention en m'appuyant sur des propos extraits de ses voeux à l'adresse de l'Union française, qu'il prononça le 22 décembre 1954 : « La Patrie, c'est tout à la fois les provinces d'outre-mer et les provinces métropolitaines, où reposent tant de nos frères morts dans les combats pour la libération des hommes. » Aujourd'hui et depuis quelques années, nous déplorons l'oubli croissant de ces combats, qui firent pourtant l'unité de notre nation, voilà encore quelques décennies. à l'approche des échéances électorales à venir, je souhaite que chacun s'en souvienne et ne nourrisse pas les populismes les plus nauséabonds, qui contribuent à désunir nos concitoyens, lesquels, j'en suis convaincu, gardent toujours en commun les valeurs de notre République

Jasmin. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je lance un appel à la paix, un véritable appel à la paix, à la suite des violences auxquelles sont confrontées les populations de la Guadeloupe, de la Martinique et, peut-être encore, de la Guyane. Les territoires d'outre-mer, en dépit de leur grande diversité géographique et institutionnelle, sont tous confrontés à des problématiques économiques, sanitaires et sociales liées à la non-adaptation de certaines politiques publiques à leurs spécificités, notamment celle de l'insularité. Ainsi, plus de dix ans après les mobilisations sociales contre la vie chère aux Antilles, nos territoires traversent de nouveau une crise sociale accentuée par la pandémie de la covid-19. En réalité, ces crises à répétition sont les conséquences des difficultés structurelles auxquelles doivent faire face ces territoires et leurs habitants.

la structuration de l'offre de formation. L'orientation et la formation professionnelle sont des enjeux majeurs pour nos jeunes et doivent donc être organisées d'urgence, afin de redonner à ceux-ci des perspectives d'avenir. Au Au préalable, un état des lieux doit être organisé pour répondre aux besoins du territoire. Je pense à la valorisation des formations et des métiers agricoles, en donnant des moyens aux lycées agricoles, pour susciter des vocations et permettre le développement de l'agrotransformation et de la diversification agricole, tout en relançant l'activité économique et touristique.

sont difficiles à vivre et le retour des natifs de nos pays est devenu une priorité. En effet, on constate un manque d'encadrement structurant pour l'émergence d'entreprises pérennes. Nos jeunes ont du talent, parfois beaucoup de talent. Ils sont porteurs de projets, mais peinent à les réaliser, faute d'accompagnement structurant. les accompagner aussi dans ce domaine, afin qu'ils puissent créer leur entreprise. Par ailleurs, aux Antilles, le chômage est endémique. Environ un jeune sur deux est au chômage et, parmi les jeunes de moins de 25 ans, le taux de chômage est de 60 %. Notons également les inégalités sociales systémiques, ainsi que la pauvreté.

de l'Hexagone. Près de 30 % des habitants des territoires d'outre-mer vivent avec moins de 850 euros par mois. En Guadeloupe, environ 135 000 personnes sont considérées comme étant pauvres. Les prestations sociales représentent 60 % des revenus des personnes les plus modestes, contre 31 % dans l'Hexagone. Une grande partie

il paraît urgent, compte tenu de la situation des territoires d'outre-mer et des impacts de la crise de la covid-19, de réguler les prix, en appliquant la loi relative à la régulation économique outre-mer.

ce qui fait considérablement augmenter les tarifs, donc les prix à la consommation ? En Guadeloupe, sur mon territoire, des questions tout aussi fondamentales- financements des travaux d'investissements sur les réseaux d'eau potable, organisation des branches professionnelles, réforme de la fiscalité des collectivités locales -doivent être abordées urgemment

Les effets de la pandémie sont dramatiques du point de vue social, d'autant que les taux de chômage et de pauvreté sont déjà, dans ces territoires, beaucoup plus élevés que dans l'Hexagone. Les effets de la pandémie sont également dévastateurs sur les économies, qui sont très dépendantes de certains secteurs, dont le tourisme, où les entreprises ultramarines sont pour la plupart des TPE. Ainsi le tourisme représente-t-il en moyenne 10 % du PIB des outre-mer. Véritable catalyseur des secteurs des transports et du commerce, il a subi un coup d'arrêt désastreux en raison de la fermeture des frontières l'an dernier.

Le tissu entrepreneurial est en très grande majorité composé de TPE, dont 70 % à 75 % d'entreprises unipersonnelles. D'un faible niveau de rentabilité, il n'est pas en mesure d'amortir le choc du confinement.

L'aggravation par la crise sanitaire de ces fragilités préexistantes compromet toute capacité à rebondir de façon rapide et pérenne dans les territoires ultramarins. Cette situation nous inquiète fortement ; elle appelle un soutien d'ampleur jusqu'à la fin de la crise, et même au-delà. Évidemment, depuis le début de la pandémie, l'État a joué et continue de jouer un rôle prépondérant et salutaire dans le soutien apporté aux économies d'outre-mer. Dès mars 2020, des dispositifs de soutien aux acteurs économiques, mais aussi aux collectivités, ont été déployés, évitant d'innombrables faillites qui auraient provoqué des dégâts irrémédiables. Les entreprises des départements et régions d'outre-mer bénéficient des dispositifs instaurés dans l'Hexagone, comme le report ou, pour les entreprises des secteurs les plus touchés,

Je souhaite que cette approche, qui tient compte des particularités locales, puisse continuer de prévaloir. Monsieur le ministre, la crise sanitaire a mis en lumière la fragilité des territoires ultramarins. Aussi apparaît-il urgent et vital d'accompagner durablement la transformation des économies dans les outre-mer, car ces territoires de la République constituent de réels atouts à valoriser. Quelles mesures le Gouvernement entend-il engager en faveur d'une véritable transformation de nos territoires ultramarins, qui sont parmi les plus pauvres de France- je pense surtout à la Guyane et à Mayotte Mayotte ? Quelles dispositions plus spécifiques envisagez-vous de prendre en faveur du logement ultramarin ? Économiquement, le BTP, secteur primordial pour les outre-mer, s'écroule dans certains territoires, comme à La Réunion.

De mon expérience d'élue locale, je conserve en effet un attachement à oeuvrer pour la prise en compte des réalités du terrain et des attentes et besoins des habitants. Prendre la parole aujourd'hui dans cet hémicycle, c'est donc l'occasion pour nous,

aucun texte spécifique aux outre-mer n'est venu changer la vie des Ultramarins ces dernières années. Nous nous attachons donc à résorber certaines inégalités par le biais d'amendements.

Pourquoi nous imposer des mesures hexagonales qui nous sont structurellement inadaptées ? Pourquoi ce qui est possible dans l'Hexagone ne l'est-il pas chez nous ? Je vous livre ici deux exemples saisissants que j'évoquerai rapidement. Le premier concerne une injustice que j'ai tenté de corriger en déposant un amendement au

les efforts déployés par nos collectivités pour réduire l'enfouissement des déchets de 80 % à l'horizon de 2025. L'un des sujets majeurs sur lesquels je souhaite aujourd'hui insister est le vieillissement de la population ultramarine, les questions fondamentales de la prévention et des conditions de logement

Là encore, nos amendements ont été rejetés, dans l'attente d'un grand plan de réforme des retraites. La solidarité familiale et intergénérationnelle a toujours été une marque de fabrique de la société domienne,

Si nos seniors sont majoritairement propriétaires, ils vivent souvent dans des logements précaires et peu adaptés à la perte d'autonomie. Une enquête réalisée voilà quatre ans démontrait de surcroît que plus de la moitié de ces logements nécessitaient des travaux. Mais le fait le plus marquant à La Réunion, par exemple, est que la dépendance s'avère toujours plus lourde et plus précoce. Il est donc impératif de mettre l'accent sur la prévention de la perte d'autonomie et d'envisager un meilleur accompagnement. Nous devons travailler au bien vieillir de nos, sur

Pourtant, cet amendement fut rejeté en séance au Sénat, le Gouvernement expliquant que la disposition proposée avait plutôt vocation à figurer dans le projet de loi relatif au grand âge et à l'autonomie, texte qui ne sera finalement jamais inscrit à l'ordre du jour du Parlement

nationale, venant mettre fin à une révolte populaire est pour le moins désastreuse. Si la politique vaccinale est indispensable, j'ai déjà exprimé mes inquiétudes, ici même, à cette tribune, quant au fait qu'elle soit guidée par la contrainte plutôt que par la conviction.

Monsieur le ministre, au lieu de la « main ferme » de l'État, c'est de la souplesse qu'il faudrait proposer. Comme l'écrivait Jean Giono : « La vie c'est de l'eau. Si vous mollissez le creux de la main, vous la gardez. Si vous serrez les poings, vous la perdez. » est d'ailleurs, avec le coût de la vie et l'affaiblissement des services publics, au premier rang desquels l'hôpital, au coeur des revendications qui s'expriment dans la rue.

Comment imaginer, dans la septième puissance économique mondiale, des robinets à sec ou déversant une eau blanche saumâtre ? Comment imaginer un rationnement tel que, depuis quatre ans, chaque commune de Guadeloupe est privée d'eau un à deux jours par semaine

Ce constat est sidérant. Il en faudrait infiniment moins, dans l'Hexagone, pour mettre les ronds-points à feu et à sang. Ce constat, vous le connaissez, bien sûr : le réseau de canalisations est vétuste et mal entretenu, ce qui entraîne une invraisemblable déperdition de 60 % à 80 % de l'eau captée 70 % des stations d'épuration sont mal entretenues, mal surveillées, et les réseaux d'assainissement privés ne sont évidemment pas aux normes. Cette catastrophe sociale se double naturellement d'une catastrophe écologique. Avec de telles pertes en ligne, le captage d'eau douce est très nettement supérieur aux besoins. Résultat : le débit des rivières diminue dangereusement, ce qui menace la continuité écologique et des pans entiers de la biodiversité de l'île. Les nappes phréatiques, souvent contaminées au chlordécone, risquent en outre la salinisation. De l'autre côté du cycle, les rejets non contrôlés et les failles béantes du système d'épuration entretiennent ou aggravent la pollution des cours d'eau et des eaux littorales. Ainsi, la pêche est interdite en Martinique dans de nombreux cours d'eau à cause du chlordécone, et les récifs coralliens souffrent grandement. L'ARS donne l'alerte : à ce rythme, à ce rythme, d'ici dix ans, il n'y aura plus de coins de baignade de grande qualité en Guadeloupe. Un désastre écologique, touristique, donc économique, est en germe. Le cas de la Guadeloupe est symptomatique ; mais j'aurais pu évoquer aussi bien les eaux contaminées au nickel, en Nouvelle-Calédonie,

insoumise, un litre d'eau sur deux est gaspillé, outre-mer, dans un réseau vétuste- gabegie invraisemblable ! ... Monsieur le ministre, vous allez me répondre que vous prenez le problème à bras-le-corps. Mais, faute d'ouvrir suffisamment les vannes financières- 170 millions d'euros pour le réseau guadeloupéen, là où il en faudrait 600 voire 700 -, le Gouvernement s'est lancé dans de la plomberie administrative en créant un nouveau syndicat des eaux. Résultat des courses : vous avez promis, ce week-end, que le problème serait réglé dans ... donc, de « tours d'eau » pour les Guadeloupéens. Il faut bien sûr aller plus vite. L'eau est un bien commun de nécessité vitale. Il faut un plan Marshall de l'eau outre-mer pour en finir avec ce désastre social, économique et écologique. Financement, ingénierie, main-d'oeuvre, l'État doit suppléer les collectivités locales partout où c'est nécessaire. Il faut mettre en place une gestion publique de l'eau et cesser de confier ce commun précieux à la prédation de Veolia et consorts. Et il faudra, le rationnement passé, instaurer la gratuité des premiers mètres cubes d'eau de compenser toutes ces années de coût invraisemblable de l'eau courante pour nos compatriotes ultramarins. Il n'y a là nul cadeau, mais une dette que nous devons solder : la dette du chlordécone, la dette de l'orpaillage, la dette du nickel

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce débat sur la situation économique, sociale et sanitaire dans les outre-mer a lieu ici, au Sénat, dans un contexte de très forte tension, avec des mouvements sociaux dans les Antilles, en Martinique et en Guadeloupe, et alors que des tensions couvent également en Guyane et en Nouvelle-Calédonie, pour d'autres raisons. Cette colère sociale s'était déjà exprimée par de puissants mouvements en Guadeloupe en 2009 et en Guyane en 2017. Elle n'a trouvé aucune réponse à la hauteur des attentes.

au passé colonial, esclavagiste, bien sûr, mais aussi au passé plus récent, lorsque l'État français permettait par dérogation l'utilisation du chlordécone, cet insecticide dont la toxicité était connue depuis 1976, mais qui a été utilisé dans les bananeraies des Antilles jusqu'en 1993- au prix de la santé des travailleuses et des travailleurs de ces exploitations. Le rejet du passe sanitaire et, dans certains cas, de la vaccination ne peut se comprendre hors de cette histoire, hors de ce contexte, où l'État français se manifeste pour imposer avec dureté et sans dialogue des mesures

On peut dire la même chose au niveau social et économique. Vous n'avez apporté aucune réponse sur le fait que 30 % des Guadeloupéens n'auraient pas accès à l'eau. Rien sur le taux de chômage, de 15 % en Martinique, de 17 % en Guadeloupe. Enfin, quelles réponses sociales apporter aux 30 % de Guadeloupéens et de Martiniquais qui vivent sous le seuil de pauvreté ? Oui, ces puissants mouvements sociaux prennent aussi leurs racines dans la lutte contre la vie chère. Pourtant, vous ne dites rien sur les marges de quelques grands groupes monopolistiques qui imposent des prix plus élevés que dans l'Hexagone. Ainsi, la bouteille de gaz coûte entre 28 et 30 euros en Martinique, et le prix tourne autour de 1,80 euro en Guadeloupe. D'ailleurs, les populations ultramarines résument très bien ce système de profit et d'exploitation issu de l'histoire coloniale par le terme créole de « profitation Après avoir légiféré, il y a quelques années, sur la transparence des prix, il nous faut passer à la vitesse supérieure et légiférer à présent sur la transparence des marges, exiger de ces grands groupes qu'ils les réduisent et bloquer les prix sur les produits de première nécessité. Enfin, les Antillais ne demandent pas autre chose que le respect et le dialogue. C'est ce que j'ai entendu la semaine dernière lors du déplacement en Guyane et en Guadeloupe que j'ai effectué Oui, il faut ouvrir le dialogue avec les élus et celles et ceux qui sont mobilisés sur la question sanitaire et la vaccination, sans contraindre, mais en tentant de convaincre. En effet, la question est complexe, mais, quand la défiance a atteint un tel niveau, la seule voie possible est le dialogue. Tout au contraire, fidèle à une trop longue tradition de l'État français, oscillant entre abandon, mépris, mensonges et promesses non tenues, vous avez choisi la voie de la fermeté et de la répression.

monsieur le ministre, ces quelques pillages et ces violences insupportables avec les femmes et les hommes, françaises et français, qui exigent l'égalité républicaine et qui sont la très grande majorité. Vous avez choisi de culpabiliser les manifestants en menaçant la population de largage politique. Un débat sur l'autonomie de la Guadeloupe ? Vous savez parfaitement que toute évolution statutaire et institutionnelle doit se faire en consultant la population : il suffit de relire notre Constitution. Cela vous permet surtout d'éviter le débat sur la question sociale. Pourtant, si vous ne savez pas par où commencer, vous n'avez qu'à lire la plateforme des 32 revendications portées par les syndicats. Je terminerai mon propos par ces quelques mots d'un des pères de la négritude, Aimé Césaire Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. » Monsieur le ministre, ne fermons plus les yeux. Réglons les problèmes de fond

en responsabilité. Alors il faut reprendre le dialogue sur place et régler toutes ces questions, pour que l'égalité républicaine résonne partout, enfin, sur l'ensemble des territoires,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je devais avoir 8 ans ou 9 ans quand, pour Noël, mes parents m'ont offert un atlas. Dans nos milieux populaires de la montagne tarnaise, c'était une période où l'on voyageait peu. Ainsi, j'ai pu voyager grâce aux cartes,

mais, quand l'État ne donne pas un bon signal en la matière, cela suscite un certain nombre d'interrogations sur bien d'autres points. Il y a la question de la jeunesse.

situation est tout simplement invivable : personne ne supporterait dans l'Hexagone ce qu'endurent nos compatriotes ultramarins dans ces deux départements.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la situation sanitaire reste évidemment un déterminant majeur de l'évolution générale des territoires ultramarins. La vague de l'été dernier, due au variant delta, y a été particulièrement violente. Certes, tous les territoires n'ont pas vécu la même détérioration sanitaire. Ceux qui les mieux protégés par un taux élevé de vaccination ont franchi cette vague sans désastre. Mais, au total, nos compatriotes ultramarins, qui représentent 4 % de la population, comptent pour 30 % des décès du pays durant cette vague. C'est insupportable À la Martinique, en Guadeloupe, en Polynésie, les morts se sont comptés par centaines. Les hôpitaux ont subi un débordement bien supérieur à celui de la première vague en métropole et les soignants ont été contraints de procéder à des priorisations de soins chez des sujets de plus en plus jeunes, âgés de moins de 50 ans. Partout, la situation est actuellement plus favorable, mais nous sommes particulièrement inquiets, car, dans plusieurs territoires, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, le taux de protection de la population par la vaccination reste bas, beaucoup trop bas.

nous appelons à accentuer la mobilisation pour la vaccination, avec le concours de relais locaux et en prenant en compte les spécificités des populations concernées. La survenue de la cinquième vague doit être anticipée par la reprise de renforts en soignants et par le renforcement de la coordination entre autorités sanitaires, établissements hospitaliers et professionnels libéraux. Les stocks d'équipements, de matériels et de produits de santé doivent être l'objet d'une attention particulière. S'agissant de l'offre de soins, les investissements en outre-mer, notamment liés au Ségur de la santé, doivent être accélérés. Pour nous, les caractéristiques géographiques et populationnelles des territoires ultramarins justifient que l'offre hospitalière soit portée, dans certains cas, au-delà des moyennes observées Enfin, la crise sanitaire met à mal l'offre générale de soins dans plusieurs territoires. Alors que celle-ci avait progressé depuis dix ans à la Réunion, en Martinique, en Guyane et en Guadeloupe, nous redoutons que l'épuisement dû à la crise et les tensions sociales et politiques qui se sont développées ne compromettent l'attractivité médicale de ces territoires. Nous appelons donc à préparer dès maintenant une stratégie pour renforcer cette attractivité. Plus que jamais, en effet, nous sommes déterminés à défendre le droit des populations d'outre-mer à accéder au même niveau de soins

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la crise de la covid-19 a durement frappé la France et le monde depuis deux ans. Elle n'est pas terminée, mais son bilan humain et social est déjà lourd. Toutefois, ses conséquences ne sont pas limitées au seul domaine de la santé publique. Elles ont pu se révéler particulièrement redoutables dans certains territoires fragiles. C'est le cas des nombreuses collectivités ultramarines, qui souffrent de problèmes économiques et sociaux profonds un taux de chômage important, notamment chez les jeunes, une forte dépendance des circuits économiques, un coût de la vie élevé, l'insuffisance de certains services publics, un manque de confiance dans les institutions. Les constats ne manquent pas pas ! Récemment, la commission des lois du Sénat a étudié une proposition de loi dont l'objectif était de rénover le service public de l'eau en Guadeloupe. Ces problématiques ne sont pas nouvelles, monsieur le ministre, et la crise sanitaire n'a fait que les renforcer. Le débat d'aujourd'hui prend tout son sens au regard des événements récents, que nul n'ignore ici. Un mouvement social important s'est déclenché en Guadeloupe et en Martinique, dépassant rapidement la question de la vaccination des soignants, Ce mouvement s'est malheureusement accompagné d'actes de violence et de destruction, que nous devons collectivement condamner- et je voudrais ici rendre hommage aux forces de l'ordre engagées outre-mer pour restaurer le calme et la tranquillité. Lors de votre très récent déplacement en Martinique, monsieur le ministre, vous avez laissé entrevoir une possibilité d'adaptation de l'obligation vaccinale. Pouvez-vous nous préciser si cette adaptation s'imposera après la date du 31 décembre, qui est celle du report de l'obligation vaccinale ? Dans ce contexte, nos outre-mer ont besoin d'un engagement ferme de la part des pouvoirs publics. Cet engagement doit se traduire au niveau national par une véritable vision pour la France d'outre-mer, prévoyant l'indispensable renforcement de la compétitivité des économies de ces territoires, ainsi que de leurs liens avec leur environnement régional. Il est essentiel, aussi, de renforcer la sécurité publique outre-mer, pour éviter la répétition des scènes de violence qui nous ont tant choqués ces derniers jours. Interrogeons-nous aussi sur la méthode à employer. Au Sénat, chambre des territoires, écho des collectivités territoriales, notre ambition doit être de passer par les collectivités ultramarines elles-mêmes, car un pilotage depuis Paris serait une nouvelle fois incompris et inefficace. Plutôt que d'ouvrir à la va-vite un débat sur l'autonomie, il serait peut-être plus sage de s'appuyer avec bon sens sur les travaux du Sénat en matière de décentralisation et de différenciation.

Après tout, ce sont bien les départements et les régions qui assument les politiques sociales et économiques. Ouvrir la voie à des statuts sur mesure permettrait aux collectivités ultramarines de disposer de marges de manoeuvre renforcées, en particulier pour adapter les normes nationales aux réalités locales. C'est ce que je dis ! Un tel statut serait la première pierre de la différenciation, car, comme vous le savez, il n'y a pas un outre-mer, mais des outre-mer. Prévoir le vote annuel d'une loi d'actualisation du droit d'outre-mer faciliterait la mise en oeuvre des politiques locales tant par les élus ultramarins que par les administrations déconcentrées de l'État, et cela assurerait le lien et la cohérence entre les politiques publiques et les spécificités locales. Par ailleurs, afin de répondre à la crise avant qu'elle n'ait lieu, il est temps de disposer d'une meilleure courroie de transmission entre les collectivités ultramarines et le Gouvernement, notamment lorsque les premières souhaitent formuler des propositions de modifications législatives. Il y a donc beaucoup à faire, monsieur le ministre, dans cette France tout entière, riche de ses territoires ultramarins. Les problématiques structurelles concernant nombre de territoires ultramarins sont restées largement les mêmes durant le mandat. Elles devront être traitées tôt ou tard afin de rétablir aussi la confiance, avant que celle-ci ne soit

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'imagine que nous sommes nombreux à nous être posé les mêmes questions devant les images des violences que nous avons vues la semaine dernière en Guadeloupe et en Martinique. telles scènes ont-elles réellement eu lieu en France ? Comment est-ce possible ? Comment a-t-on pu en arriver là ? Ce qui s'est passé ces derniers jours dans les Antilles semble tout bonnement impensable, mais ces événements ont bel et bien eu lieu. Ils sont symptomatiques d'une crise aux racines bien plus profondes qu'une contestation de l'obligation vaccinale des soignants et du passe sanitaire. La crise qui se manifeste aujourd'hui dans les outre-mer est complexe. Elle est multiface et à plusieurs degrés, du plus urgent au plus profond. La priorité qui devait être la nôtre était la sécurité. Il était urgent de rétablir l'ordre et de faire preuve de force et de fermeté face aux violences. Si les revendications des populations d'outre-mer sont légitimes, de telles actions étaient tout simplement inacceptables, et il devait y être mis fin au plus vite. Les tensions se sont désormais calmées et l'envoi de policiers et de militaires supplémentaires était bienvenu. Mais je ne peux que regretter que cette décision ait pris tant de temps à intervenir. Je souhaite désormais que la justice fasse preuve de la plus grande fermeté envers les auteurs de telles exactions, en particulier envers ceux qui se sont rendus coupables de violences sur les forces de l'ordre. Il est de notre devoir d'être intransigeants à cet égard. La deuxième problématique qui doit être au centre de nos préoccupations a trait à la situation sanitaire. L'obligation vaccinale pour les soignants et le passe sanitaire sont, en surface, les raisons qui ont précipité les outre-mer dans une telle crise. Alors que près de 80 % de la population est vaccinée dans l'Hexagone, le taux de vaccination le plus élevé en outre-mer est de 60 % pour La Réunion et le plus bas n'atteint même pas 23 % en Guyane. Ces disparités doivent conduire à nous interroger et à nous adapter. Elles mettent en lumière une réelle absence de confiance des populations envers le pouvoir central et ses décisions, ainsi qu'en la médecine. Les récentes décisions du Gouvernement visant à repousser l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale et à prioriser les vaccins sans ARN pour les outre-mer étaient nécessaires, mais elles ne suffiront pas. Des mesures fortes devront être prises pour retisser les liens de confiance, qui- soyons honnêtes -ne sont plus là depuis de nombreuses années.

Ce droit existe ; il faut l'appliquer. Au lieu de désengager l'État des outre-mer, nous devons au contraire l'y renforcer, réinvestir dans ces territoires et les accompagner tout en veillant à ce que celui-ci respecte leurs spécificités et s'y adapte.

La date du scrutin a été maintenue, la situation épidémique étant désormais sous contrôle, mais elle continue de faire l'objet de trop nombreuses polémiques. Elle a pourtant été soutenue par des personnalités de la société civile appelant à mettre fin à l'incertitude institutionnelle, qui n'a- nous en sommes tous convaincus -que trop duré. Après deux précédentes consultations ayant confirmé la volonté du peuple calédonien de demeurer dans la République, cette dernière consultation optionnelle sera- j'en suis sûr -l'occasion de sortir d'une telle impasse et d'éviter une surenchère. Je tiens à réaffirmer ma volonté que la consultation aille à son terme dans les meilleures conditions et qu'elle permette d'ouvrir une nouvelle page, un nouveau contrat social, entre la métropole et le Caillou. Car la métropole n'a jamais laissé de côté la Nouvelle-Calédonie. de juin 1988, la paix et l'exercice pacifique du droit à l'indépendance ont éclipsé la violence et l'incompréhension. Au mois de septembre dernier, une centaine de réservistes sanitaires ont été envoyés pour aider la population. En 2021, quelque 178 milliards de francs CFP ont été investis par l'État pour la Nouvelle-Calédonie, partagés notamment entre les dépenses d'intervention et l'aide fiscale à l'investissement. Dès lors, monsieur le ministre, comment abordez-vous ce scrutin aussi stratégique que détourné de son objectif véritable ? Comment ouvrir une nouvelle page dans la relation entre la France et la Nouvelle-Calédonie ? La parole est à M. le ministre. Monsieur le sénateur

La mise en berne des activités économiques à la suite du confinement et des mesures de restrictions sanitaires ont exacerbé les faiblesses structurelles du tissu entrepreneurial ultramarin, majoritairement composé de petites entreprises et fortement dépendant du tourisme. Je rappelle que, pour tenter d'endiguer la crise, le Gouvernement a étendu dans les outre-mer les dispositifs de soutien que sont le fonds de solidarité pour les entreprises ou encore les prêts garantis par l'État. Or j'attire votre attention, monsieur le ministre, sur un point jusqu'ici peu évoqué : si l'impact des premières vagues épidémiques a été généralement moindre dans les outre-mer qu'en métropole, ces derniers subissent aujourd'hui de plein fouet la double crise sanitaire et économique. Il est donc urgent, et même vital, de synchroniser les dispositifs d'aide économique aux outre-mer, de ce décalage de l'épidémie dans le temps. Monsieur le ministre, puisque les mesures économiques ont précédé l'explosion de la pandémie dans les outre-mer, comptez-vous réadapter rapidement ces dernières à la crise actuelle ?

je souhaitais saisir l'occasion de ce débat pour clarifier un peu les choses et nous permettre, collectivement, d'avancer à la suite de votre déplacement. « Nous ne serons jamais de ceux qui contestent votre fermeté face aux demandes d'amnistie des délinquants, pas plus que votre volonté de rétablir l'ordre. Pour autant, nous considérons que le choix délibéré d'une visite express, à la symbolique militaire et à la posture martiale et autoritariste, est une grave erreur politique. « Vous ne pouvez ignorer que cela a braqué, a choqué et surtout- c'est là le plus grave -légitimé l'action politique de ceux qui, de toute façon, ne sont pas là pour discuter. « Il était tout aussi maladroit de prétendre que tous les problèmes de l'île relèvent uniquement de compétences locales. Cette défausse ne pouvait que tendre le dialogue, y compris avec vos alliés politiques locaux et membres de votre majorité. définitive, par ses excès, ce malheureux épisode n'a fait que renforcer la stratégie de pourrissement voulue par certains. « Dans le même temps, et bien que vilipendés et délégitimés, les élus prennent leurs responsabilités en écoutant et en proposant. À l'État désormais de prendre les siennes. « Monsieur le ministre, dans avec quels experts, quels collègues et surtout avec quelle volonté reviendrez-vous en Guadeloupe pour non pas renouer, mais bel et bien nouer le dialogue et ainsi éviter la montée aux extrêmes et les morts ? « Cette crise ne doit pas devenir une occasion d'envenimer le climat pour plaire à une frange radicalisée de l'opinion publique hexagonale

il y a quelques jours, la Guadeloupe et la Martinique s'embrasaient et connaissaient des scènes d'insurrection inquiétantes et désolantes. À la faveur de votre déplacement, vous avez pu personnellement évaluer la situation sur le terrain. Les revendications de ces agitateurs et casseurs, chauffés à blanc par certains syndicats aussi, ne paraissent pas, hélas, clairement identifiées. Il n'en reste pas moins que ces violences sont intolérables. Comme dans les autres territoires d'outre-mer, le gouvernement français a fait de gros efforts sur les plans de la vaccination et de la protection sanitaire.

Pourtant, tout est bon en termes de récupération politique pour jeter de l'huile sur le feu. La pseudo-polémique entraînée par vos propos sur une plus grande autonomie de la Guadeloupe semble davantage liée à des tensions politiques de période présidentielle qu'au tabou de l'autonomie, qui n'a pas lieu d'être dans notre cadre constitutionnel. Monsieur le ministre, pensez-vous que les discussions et les échanges que vous avez eus avec des responsables politiques locaux puissent ramener un peu de calme et de sérénité sur ces deux îles ? Voyez-vous d'autres solutions pour sortir de cette crise ?

à ces territoires de trouver les conditions d'un développement harmonieux et d'une croissance économique permettant de lutter efficacement contre le chômage, en particulier celui des jeunes. Il faut agir de concert sur l'emploi et sur la consommation des ménages, afin de créer un choc de revitalisation économique. Il y a, outre-mer, un véritable problème de coût du travail : son niveau élevé, en comparaison des territoires voisins, limite la compétitivité des entreprises locales. Il est pourtant nécessaire de permettre à ces entreprises de développer leurs activités, d'investir, d'innover, de baisser leurs prix et de recruter des collaborateurs.

la presse, il y a quelques jours. Dans ces conditions, ne devrait-on pas favoriser l'insertion dans les entreprises du secteur privé ? Quelle est la stratégie du Gouvernement pour développer les entreprises ? Dans le cadre du grand débat national,

la Guyane a traversé une crise sanitaire sans précédent, qui a mis les personnels des trois seuls hôpitaux guyanais au bord de la rupture. Ces derniers mois, alors que le taux d'incidence frôlait les 500 cas pour 100 000 habitants,

Quand, à ces inégalités d'accès aux soins se conjuguent- cela a été dit -vie chère, un taux de pauvreté à près de 53 % et un revenu médian d'à peine 900 euros ? Les Antilles s'enflamment pour les mêmes raisons : ces inégalités sociales et sanitaires territoriales qui perdurent,

L'obligation vaccinale des soignants et des pompiers a mis le feu aux poudres dans un contexte multidimensionnel devenu insupportable pour nos outre-mer. Mon camarade Fabien Gay et d'autres collègues ont multiplié les exemples de ces inégalités vécues et subies

Nos compatriotes ultramarins manifestent aujourd'hui pour une revalorisation de leur pouvoir d'achat, pour une progression des salaires, pour des moyens de sortir de la précarité, etc. Ils manifestent tout simplement pour plus d'égalité et pour vivre dignement ! Comme l'a dit Fabien Gay, nous condamnons avec fermeté toutes les violences,

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, si nous nous interrogeons aujourd'hui sur les politiques à mener pour l'éducation et la jeunesse, c'est bien parce que nous ressentons un malaise dans ce domaine. Est-ce que l'éducation de la jeunesse est perçue comme la priorité dans notre société ? Dans un monde de perpétuelle indignation, de revendications de droits individuels, avons-nous gardé comme priorité le devoir collectif d'éduquer notre jeunesse ? Un de mes grands regrets pour l'année 2020 est que nous n'ayons pas pu fêter dignement le 150 anniversaire de la République et en tirer les enseignements. Cette III République

Et la République radicale, en faisant de l'éducation sa priorité avec l'école publique, laïque, gratuite et obligatoire, en formant une élite de la Nation, ces hussards noirs de la République envoyés dans chaque village et école, a su faire de la France, en une génération, un pays qui était en 1900 à l'avant-garde dans l'automobile, l'aviation, la chimie ou le cinéma ... Nous avons le même défi à relever aujourd'hui : voulons-nous vraiment faire à notre tour de la jeunesse et de l'éducation notre priorité ? La richesse de notre pays est sa ressource humaine : le travail et l'intelligence de nos concitoyens. Alors, investissons, comme toute société responsable, dans notre production de richesse, dans nos ressources humaines, dans notre jeunesse. Le constat est consternant

Devant le constat de tous ces manques, que proposons-nous ? On compense le manque d'activité physique par un Pass'Sport, le manque d'accès à la culture par un pass Culture, le manque d'esprit civique par un service national universel, etc. Autant de petits pansements sur une plaie trop béante

Certaines écoles proposent d'ailleurs de réaliser le deuxième cycle du second degré en quatre ans avec l'acquisition d'un CAP, d'un BEP ou du baccalauréat. Autant d'innovations qui permettent à certains jeunes de toucher de la matière et de se structurer pour s'ouvrir à d'autres horizons. On peut s'interroger aujourd'hui sur la nécessité d'une année supplémentaire à l'issue du secondaire afin de compléter l'enseignement par les notions de civisme, de laïcité, de secourisme, mais aussi par le code de la route pour combler cette grande injustice d'un permis de conduire trop cher pour certaines familles.

madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, les difficultés de la jeunesse ont été cruellement dévoilées par les effets de la crise sanitaire sur les plus précaires des 18-25 ans. Dans son portrait social de la France publié le 25 novembre dernier, l'Insee souligne par exemple que la prévalence des syndromes dépressifs chez les 18-29 ans a fortement augmenté, alors qu'elle est restée stable au sein des autres classes d'âge. Dans un autre registre, en 2020, le taux d'emploi des 18-24 ans a baissé de 1,7 point par rapport à 2019, alors qu'il est resté stable pour les 30-64 ans. Les problèmes rencontrés par la jeunesse sont cependant incontestablement plus anciens. Pour mémoire, dans son rapport annuel de 2020 sur l'état de la pauvreté en France intitulé, le Secours catholique le Secours catholique confirmait la situation de crise profonde que traversait la jeunesse dès avant la crise de la covid-19, en rappelant par exemple que les niveaux de vie des deux tranches d'âge 15-24 ans et 25-34 ans se situent largement sous le seuil de pauvreté : 139 euros pour les premiers et 413 euros pour les seconds. Ces constats, qui témoignent d'une inégalité des chances et des droits qui pénalise de trop nombreux jeunes, ont conduit le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain à défendre la proposition de loi relative aux droits nouveaux dès 18 ans et à demander l'installation d'une mission d'information sur la politique en faveur de l'égalité des chances et de l'émancipation de la jeunesse, dont j'ai été la rapporteure. Au fil des travaux menés dans le cadre de cette mission, il est apparu que les difficultés rencontrées par la jeunesse se déclinent sur tous les plans, de la formation à la santé, en passant par l'accès à l'emploi et à la culture. La nécessité de penser l'accompagnement de la petite enfance à l'âge adulte s'est également imposée. Le développement du jeune enfant et les acquis intervenus au cours des toutes premières années ont en effet des incidences sur ses compétences et sa santé futures. Les inégalités se forment dès ce stade. À l'autre extrémité du spectre, concernant les jeunes adultes, nous savons que la France compte environ un million de « NEET », des jeunes sortis du système scolaire, mais qui ne sont ni en emploi ni en formation. Ils sont plus de deux millions, en englobant les jeunes ayant suivi des formations ou exercé des activités sur un temps réduit- ils connaissent également des situations de forte précarité. Chaque public doit être accompagné en prenant en compte son environnement afin de permettre à chacun de bénéficier des meilleures chances et du plein respect de ses droits. Pour répondre à ces besoins, un ensemble hétérogène et foisonnant de dispositifs existent, mais ils sont, pour une majeure partie d'entre eux, difficilement identifiés aussi bien par les jeunes et leurs familles que par certains acteurs. Les politiques en faveur de la jeunesse et de l'égalité des chances touchent de fait à de nombreux domaines de l'action publique. Elles mobilisent des acteurs nationaux et locaux très variés : État, collectivités territoriales, organismes publics et privés. Alors que certaines pistes sont négligées, telles que l'éducation populaire qui offre pourtant une éducation hors milieu familial et scolaire porteuse d'autonomie et d'émancipation, l'existant est très intéressant, mais ne fait l'objet ni d'une politique suivie, ni d'une évaluation, ni d'investissements suffisants. Les conclusions du rapport de la mission d'information sur la politique en faveur de l'égalité des chances et de l'émancipation de la jeunesse insistent donc sur la simplification, la valorisation et la mise en cohérence de ce qui est déjà mis en oeuvre. Par ailleurs, à l'occasion des auditions menées dans le cadre de cette mission d'information, l'immense majorité des personnes et structures entendues ont pris position en faveur d'un revenu de subsistance pour les moins de 25 ans, quelle que soit sa forme.

de manière dégressive en fonction des revenus de la personne, pour garder une réelle incitation au travail, et de manière inconditionnelle, pour permettre aux travailleurs sociaux de concentrer leurs interventions sur l'accompagnement et non sur le contrôle des personnes. Par ailleurs, un dispositif de dotation universelle ouvrirait un compte personnel d'activité pour toute personne à ses 18 ans avec un crédit de 5 000 euros librement utilisable pour des projets de formation, de mobilité ou d'entrepreneuriat. Le revenu de base inconditionnel et la dotation universelle seraient financés par une fiscalité plus juste des hauts patrimoines, des hauts revenus et des multinationales. Les jeunes doivent avoir accès aux mêmes droits que les plus anciens.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, l'école est cet espace d'élévation dans lequel l'enfance dessine l'avenir et le fait advenir. Parce qu'elle est un moment charnière dans l'existence, nous devons tout faire pour offrir aux enfants cet héritage indispensable que forme l'éducation dans l'esprit de chacun. Investir massivement dans l'école, dès le plus jeune âge, voilà la priorité ! Ces dernières années, le Gouvernement a concentré ses moyens en direction des publics identifiés comme les plus fragiles, en dédoublant progressivement les classes de grande section de maternelle, de CP et de CE1 des réseaux d'éducation prioritaire Ces mesures semblent porter leurs fruits : les études constatent dans ces classes une amélioration du climat scolaire et de meilleurs résultats, en particulier en mathématiques. Nous y sommes favorables dans la mesure où elles contribuent à lutter contre le déterminisme social, en offrant de meilleures conditions d'apprentissage aux élèves qui en ont le plus besoin. Pourtant, nous devons changer d'échelle, aller plus loin, plus haut, dirai-je. Le Gouvernement entend limiter progressivement les effectifs à 24 élèves par classe à l'école élémentaire, soit la moyenne actuelle. Je pense qu'il nous faut être plus ambitieux et abaisser cette jauge à 22 élèves par classe pour favoriser l'apprentissage des fondamentaux dans de bonnes conditions. Le nombre d'élèves « non lecteurs » est en augmentation, tandis que le niveau des élèves baisse continuellement depuis près de vingt ans. Très concrètement, ou un enseignant en fin de carrière ne peut plus proposer à ses élèves les mêmes exercices qu'elle ou il proposait voilà trente ans aux élèves du même niveau. Nous devons fournir plus d'efforts pour inverser la tendance et améliorer les résultats des élèves en leur donnant le goût du travail. Pour cela, aux élèves en difficulté (Rased), ce qui permettrait d'offrir un accompagnement adapté aux élèves le plus en difficulté et un soutien inestimable pour les enseignants. Nous ne devons laisser aucun élève illettré sans accompagnement ciblé scolaire (AVS) par semaine, dans une classe de CM1 de 28 élèves, dont deux enfants « non-lecteurs », voilà la réalité quotidienne de bon nombre d'enseignants à qui l'on demande des résultats sans les moyens, c'est-à-dire l'impossible. ailleurs, la faiblesse des évaluations dites « courtes, ciblées et valorisantes », associée au nombre insuffisant d'évaluations nationales, ne permet pas un suivi régulier des acquis, des lacunes et des progrès des élèves. Si nous voulons changer de dynamique, il nous faut mettre en place des évaluations nationales standardisées à chaque étape, c'est-à-dire à chaque classe, et j'irai même plus loin : je pense que nous devons systématiquement évaluer les élèves à la rentrée et en fin d'année de chaque classe, avec un dispositif adapté aux classes multiniveaux, lesquelles concernent près d'un élève sur deux. Il suffirait pour cela de flécher 6 heures des 108 heures de réunion par an des enseignants pour corriger ces évaluations. Cette mesure permettrait de donner une vision homogène des exigences, de mettre en évidence les élèves en grande difficulté afin de renforcer leur accompagnement, et d'identifier les élèves les plus prometteurs. Nous devons guider les plus fragiles vers la réussite en prévoyant un parcours suffisamment stimulant pour les élèves que je qualifierai d'« agiles ». En effet, près d'un tiers des enfants à haut potentiel se retrouve en échec scolaire, faute d'une scolarité adaptée. Il faudrait également augmenter- pourquoi pas doubler ? -le temps consacré aux échanges individualisés avec les parents afin de permettre à chaque enseignant de rencontrer chaque parent d'élève au moins quinze minutes par an. Nous devons également accorder plus de souplesse dans le choix des 18 heures de formation annuelle des enseignants. Bien souvent, ils sont contraints de suivre des formations déconnectées de la réalité, éloignées de leurs besoins et en décalage par rapport au déroulé du programme. La plupart des enseignants ont un immense besoin de formation et de soutien dans la gestion de la classe. Ils devraient aussi pouvoir bénéficier de rendez-vous avec un psychologue scolaire tout au long de l'année, autant que de besoin.

ces grandes lignes programmatiques sont les quelques ajustements nécessaires pour que l'« âge d'or » de l'éducation nationale soit non pas derrière nous, mais droit devant.

Toutes ces mesures ont-elles eu pour autant sur notre école l'effet de revitalisation escompté ? Je vous propose de choisir deux thèmes pour le mesurer, en abordant en premier lieu le renforcement de l'enseignement des disciplines fondamentales. Le français, la morale, le calcul ! » s'exclamait Jules Ferry. Par-delà la formule, le ministre affirmait sa volonté de mener tous les citoyens au niveau d'éducation nécessaire à l'exercice de leurs responsabilités démocratiques. Forte de ce socle, l'école républicaine a progressivement nourri l'image d'une école capable d'offrir à tous la possibilité de s'élever dans la société par le travail, la motivation et le mérite. Autant de valeurs dont la remise en cause, à partir des années 1960,

a dit sa volonté de refaire de l'école élémentaire celle du « lire, écrire, compter ». Renouant avec la pratique des circulaires, il a fixé un cadre général à l'enseignement de ces fondamentaux. Pourtant, plus les enquêtes se succèdent et moins le doute est permis : les résultats de tous les élèves baissent inexorablement, même pour les meilleurs d'entre eux. Les comparaisons européennes et mondiales sont affligeantes.

Le phénomène est global et durable, mais c'est Jean-Michel Blanquer qui a dirigé le dernier le ministère de l'éducation nationale, et ce sur une durée sans équivalent depuis Victor Duruy et le Second Empire. La question est simple l'enseignement des disciplines fondamentales à l'école élémentaire a-t-il été au moins partiellement redressé ? Certes, le gouvernement auquel vous participez, madame la secrétaire d'État, a engagé un certain nombre de grands chantiers, qui vont pour la plupart dans le bon sens, comme le dédoublement des classes en REP et REP+, le plafonnement des effectifs du primaire ou la réforme de la formation initiale des professeurs. Pour autant, l'impression qui prédomine est que nous sommes encore prostrés au milieu du gué. Le « en même temps » n'a finalement abouti qu'à des demi-mesures, provoquant d'entières déceptions. Des demi-mesures qui s'avèrent bien insuffisantes pour soigner les maux d'une école qui a besoin d'une politique de franche rupture. Mais vous n'en aviez pas les moyens politiques. Sur certaines travées, on nous rejouera l'air du manque de moyens, éternel refrain qui n'a jamais réduit un tant soit peu l'affaiblissement des résultats enregistrés enquête après enquête. J'ai quant à moi l'intime conviction que seule la rupture avec une école qui a abaissé la parole du maître et la transmission des savoirs permettra de rompre avec cette tendance infernale. Parler de la parole du maître, c'est aussi s'interroger sur la place des professeurs dans la société. Sur ce point, l'échec de ces dernières décennies est tout aussi retentissant. Dans le pays où Victor Hugo qualifiait les maîtres d'école de « jardiniers en intelligence humaine », seuls 7 % des professeurs estiment que leur profession est appréciée. Alors que 364 professeurs démissionnaient en 2008, ils sont près de 1 500 à déserter aujourd'hui le « professeur » et la violence exercée par les parents, même parfois par les élèves. Jadis piliers de la République, ils ressentent désormais un sentiment d'abandon. Certes, le Grenelle de l'éducation est un début de prise en considération, mais, au-delà, ils attendent surtout d'être soutenus quand leur autorité soutenus quand leur autorité est contestée. Or l'on continue de les culpabiliser, en leur disant, par exemple, qu'ils ne sont pas capables d'appréhender la diversité des élèves d'aujourd'hui. Et si la solution consistait plutôt, pour une fois, à leur faire confiance et à laisser des espaces de liberté à ces praticiens de terrain que sont les proviseurs, les principaux et les professeurs Or le ministère Blanquer n'aura pas été celui d'une plus grande liberté pour les équipes et d'une plus grande autonomie pour les établissements. Le ministre n'a pas su ou n'a pas pu desserrer l'étau étouffant du dernier système éducatif centralisé et bureaucratisé d'Europe. Pour ma part, je suis persuadé que cette école de la confiance, que Jean-Michel Blanquer appelait de ses voeux en début de quinquennat, ne pourra être construite qu'en faisant confiance et en libérant les énergies. Ainsi, l'école redeviendra le ferment de notre République.

permet de questionner un sujet central : la place de la jeunesse dans l'ensemble de nos politiques publiques. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que, dès lors que l'on appréhende ce sujet de manière globale, le constat est peu reluisant pour ce gouvernement. Que veut dire être jeune sous Emmanuel Macron ? Tout d'abord, concernant les conditions matérielles, la précarité de la jeunesse est criante. Elle s'est manifestée de façon spectaculaire dans l'espace public pendant la crise du covid-19 par ces longues files d'attente devant les banques alimentaires, mais elle n'est pas nouvelle. Dans notre pays, près de 1,5 million de jeunes sont soit travailleurs pauvres, soit ni en emploi ni en formation, et un jeune sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Pourtant, face à ce constat alarmant, le soutien financier à la jeunesse ne fait manifestement pas partie des priorités du Gouvernement. Leur accès aux droits sociaux est ainsi toujours extrêmement entravé. les jeunes sont très majoritairement privés du dispositif de l'assurance chômage. La durée de travail minimale nécessaire de 6 mois sur 24 mois pour bénéficier de l'allocation tend en effet à écarter de nombreux jeunes, qui n'ont accès qu'à des emplois courts et très précaires. et très précaires. Pis, durant le confinement, 58 % des étudiants ont été forcés d'arrêter, réduire ou changer leur activité rémunérée. Pour les étudiants, il est quasiment impossible d'accéder à l'assurance chômage, puisque celle-ci est liée à une recherche active d'emploi, considérée par Pôle emploi comme incompatible avec une scolarité universitaire. Ils travaillent, cotisent, mais n'ont droit à rien. Les jeunes n'ont pas plus accès au RSA. Toute cette partie de la population, soit les 18-25 ans, est volontairement écartée de cet indispensable amortisseur social au motif que, selon M. Bruno Le Maire, « à 18 ans, ce qu'on veut, c'est un travail, et et pas une allocation ». Cette affirmation n'est pas seulement paternaliste et méprisante ; elle est aussi un déni de réalité économique. Le ministre de l'économie devrait relire la lauréate du prix Nobel d'économie, Esther Duflo, dont l'ensemble des travaux démontrent qu'il n'y a qu'il n'y a absolument pas d'effet décourageant face au travail quand on perçoit des aides sans condition. Bien au contraire, plus on aide les gens, plus ils sont capables de repartir d'eux-mêmes, plus ils sont aptes à sortir de la pauvreté. Vous privez donc la jeunesse d'un peu de dignité économique pour des raisons purement idéologiques. Au-delà de leur niveau de vie se pose aussi la question de la santé de la jeunesse. Un tiers des étudiants déclarent avoir renoncé au moins une fois à des examens ou soins médicaux au cours de l'année 2020 pour des raisons financières. Rien d'étonnant, quand on sait qu'un tiers des jeunes ne sont toujours pas couverts par une mutuelle. Si le Gouvernement a mis en place la complémentaire santé solidaire, qui remplace la CMU-C et élargit son périmètre, la Cour des comptes note dans un rapport que les étudiants ne sont pas concernés par le renouvellement automatique de cette couverture. Ils sont ainsi obligés, chaque année, de refaire leur dossier, ce qui augmente inexorablement le taux de non-recours. Au niveau de la santé mentale, là aussi, les chiffres sont inquiétants. Un tiers des étudiants ont présenté les signes d'une détresse psychologique durant le confinement et les files d'attente devant les psychologues universitaires se sont allongées durant la pandémie. chèque psy », avec le remboursement de trois séances annuelles, a été mis en place, tardivement, par le Gouvernement, cette mesure, certes bienvenue, ne nous semble pas à la hauteur pour faire face à l'urgence. Enfin, quelles perspectives offrir à la jeunesse ? Au-delà des injonctions creuses et paternalistes sur la valeur travail, quelle mesure concrète, quelle politique emblématique pour l'avenir le Gouvernement a-t-il mise en place pour remobiliser la jeunesse ? Le service national universel (SNU) ! Ce service, qui surfe sur la nostalgie naïve du service militaire, reposant sur une vision surannée de l'ordre républicain, le petit doigt sur la couture du pantalon, et sur le fantasme d'une jeunesse en uniforme, qui apprend à saluer et marcher au pas, ne correspond à aucun enjeu ni aucune aspiration de notre époque ou de notre jeunesse. Pour autant, son budget a quasiment doublé, passant de 62 millions d'euros à 110 millions d'euros, pour un service qui n'a rien d'universel : parmi les volontaires, seuls 4 % proviennent des quartiers populaires, un chiffre à mettre en parallèle avec les 37 % de volontaires qui ont des liens familiaux avec des personnes portant l'uniforme. Le public est donc pour l'instant très spécifique. On est très loin des objectifs initiaux et son caractère universel n'est qu'une illusion. Alors que la crise a été révélatrice de la précarité et des difficultés d'accès aux droits de la jeunesse, les réponses du Gouvernement manquent complètement leur cible. À cela s'ajoute

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, ce débat doit nous permettre à la fois de tirer le bilan éducatif du dernier quinquennat et de dégager des perspectives nouvelles. Ces cinq années auront été marquées, à presque tous les niveaux de la scolarité, par un sous-investissement chronique. Oui, l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur représentent respectivement les premier et troisième budgets de l'État c'est un fait ! Oui, les crédits généraux accordés à ces deux secteurs ont crû de 8 milliards d'euros et 4 milliards d'euros, hors plan de relance. Toutefois, derrière ces chiffres se cache une autre réalité. En quinze ans, la part de l'éducation dans le PIB a reculé d'un point et est en baisse constante. Pis, la part de l'État

Face à cette situation, deux choix étaient possibles : réinvestir massivement ou gérer la pénurie. C'est malheureusement le second choix qui a été fait, avec, en prime, un chantage insupportable, en tout cas dans ma ville, à Marseille : « On vous aidera à rénover vos écoles si vous acceptez le recrutement sur profil.

comme seule condition d'accession. Parcoursup n'a fait que généraliser la problématique que nous connaissions avec le système d'admission post-bac (APB), sans pour autant ajouter de l'humain. Le ministère se targue d'un très faible nombre de recalés à l'entrée de l'université. Il est bien le seul

ainsi récemment : « Dès qu'une mesure sélective est prise chez vous, cela se ressent ici. » Cette année, le ministre va encore plus loin en instaurant le Parcoursup des masters. Bien sûr, il s'appuie sur la réforme de ses prédécesseurs, qui, eux aussi, avaient fait le choix de traiter le manque de places par la sélection, à la systématiser. Pourtant, les occupations récentes des universités de Nanterre ou de Lyon 2 montrent que le problème est non pas le niveau des étudiants, mais bien le manque de moyens accordés aux universités pour remplir leurs missions. L'institution scolaire et universitaire est aujourd'hui à bout de souffle. Elle ne tient plus que grâce à l'engagement sans faille de ses personnels. Ces derniers, fort peu soutenus par leurs ministres de tutelle, jamais avares de polémiques stériles, font aujourd'hui partie des enseignants les moins Injonctions contradictoires, stigmatisations et précarisation ont été les maîtres mots de ces cinq dernières années, au point même que les hauts fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, pourtant peu bavards en règle générale, se sont fendus non pas d'une, mais de deux tribunes publiques d'alerte. d'alerte. Ce dont a besoin aujourd'hui l'école, c'est donc d'un réinvestissement massif. À ce titre, le recrutement de 90 000 enseignants sur cinq ans, accompagné d'une réelle revalorisation des traitements, doit permettre de limiter le nombre d'enfants par classe et d'améliorer les conditions de travail des enseignants. Par ailleurs, parce que l'école doit redevenir le lieu où se gomme la reproduction des inégalités sociales, parce qu'elle doit être le lieu de l'émancipation, il faut repenser une nouvelle fois les rythmes. Le passage à 32 heures hebdomadaires d'enseignement ou de suivi pédagogique, couplé à la fin effective des devoirs à la maison, doit permettre d'atteindre cet objectif. En effet, des enfants ne pouvant pas s'appuyer sur leurs proches ou ne disposant pas de bonnes conditions matérielles pour faire leurs devoirs partent déjà avec un temps de retard. appris pour l'école doit l'être à l'école. Enfin, il faudra faire l'inventaire des réformes qui se sont succédé dans l'enseignement. Je les rappelle pêle-mêle : la sélection à l'entrée en licence et en master, la réforme du lycée et du baccalauréat, le passage à trois ans du baccalauréat professionnel, la concentration à outrance sur les savoirs fondamentaux. Le

à les creuser. Dans cette période traversée par une surenchère sécuritaire, je ne peux m'empêcher de penser à la célèbre citation de Victor Hugo : « Celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison. » Faisons donc toutes et tous ensemble le pari de l'école pour demain. La parole

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le 22 novembre dernier, le journal révélait, à sa une, le nombre grandissant des démissions d'enseignants.

l'année dernière, on ne relevait pas moins de 937 démissions dans le premier degré et 617 dans le second degré. Le nombre de ces démissions a été multiplié par trois entre 2013 et 2018

Je souhaite cependant attirer l'attention sur un facteur souvent minimisé : la mobilité des enseignants. La possibilité de choisir son lieu de travail est primordiale et souvent déterminante dans la poursuite d'une carrière professionnelle. Dans le cadre du Grenelle de l'éducation, le Gouvernement a pris l'engagement d'accompagner la mobilité des enseignants. Pourtant, la plupart d'entre eux semblent réservés et font face à des « embouteillages », selon le terme de Maxime Reppert, membre du Syndicat national des lycées, collèges, Madame la secrétaire d'État, que comptez-vous mettre en place, concrètement, pour faciliter l'exercice de la mobilité des enseignants ? Au malaise de ces derniers s'ajoute parfois celui des élèves. Le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement concernent entre 800 000 et 1 million d'enfants ; autrement dit, entre 6 % et 12 % des élèves subissent ou ont subi une forme de harcèlement au cours de leur scolarité. Aucun établissement, aucune région, aucune catégorie sociale ne sont épargnés. Face à cette réalité, le corps enseignant s'estime souvent désarmé, du fait d'un manque de formation, et souligne des difficultés à identifier les cas de harcèlement. Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire, le Président de la République a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre ce fléau, notamment la mise en place d'une application de signalement. Si toute action visant à mettre un terme aux pratiques de harcèlement scolaire doit être saluée, nous regrettons que les conclusions rendues par la mission d'information sénatoriale sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement n'aient pas encore trouvé d'écho. Ce rapport met en avant 35 recommandations concrètes pour une lutte efficace contre le harcèlement et le cyberharcèlement. Seul un enseignant sur trois s'estime armé pour lutter contre ce fléau. Il apparaît donc essentiel que les enseignants, dans le cadre de leur formation initiale, soient éduqués à la prévention des faits de harcèlement.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, depuis bientôt cinq ans, une logique implacable est à l'oeuvre en matière d'éducation : celle d'une vision libérale de l'école, en contradiction avec le modèle de l'école publique républicaine que nous chérissons. Durant ce quinquennat, il a toujours été question de faire des économies, en augmentant considérablement le recours aux contractuels et en supprimant des postes. Près Près de 8 000 postes ont ainsi été supprimés dans le secondaire depuis 2017, alors même que 25 000 élèves supplémentaires sont attendus à la rentrée 2022. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur l'enseignement agricole, dont les effectifs ont chuté de 300 postes : cela correspondrait, en proportion, à une suppression de 10 000 postes dans l'éducation nationale ! Toutes ces suppressions devaient permettre de créer des postes dans le premier degré, présenté comme une priorité absolue. Dans les faits, il n'en est pourtant rien : il n'y aura d'ailleurs aucune création de postes dans le primaire à la prochaine rentrée. Or les retours du terrain sont unanimes

à fermer des classes et à perdre des postes de remplaçants, dont le manque se fait sentir de plus en plus durement. Loin du discours affiché de rééquilibrage en faveur des classes sociales défavorisées, nous constatons que, dans l'ensemble, les réformes qui se sont enchaînées depuis 2017 s'inscrivent dans le sillon d'une logique inégalitaire. Parcoursup en est un exemple flagrant : si nous voulons lutter contre la reproduction des inégalités sociales et territoriales, qui se sont encore aggravées depuis la mise en place de cette plateforme, il faut sortir de cette logique de sélection accrue et dépersonnalisée, afin de redonner toute sa place à un processus d'orientation au plus près des besoins et des vocations des élèves. Tous les indicateurs le prouvent : il est urgent de redonner corps à la promesse républicaine au sein de notre système scolaire, il est urgent de redémarrer l'ascenseur social Cela nécessite notamment de nouvelles ambitions fortes en matière de mixité sociale et de lutte contre les ghettos scolaires. Contrairement à ce que pense le Président de la République, ce n'est pas en demandant aux directeurs et directrices d'école de recruter leur personnel comme le feraient des chefs d'entreprise que nous y parviendrons. Cela passe aussi

Enfin, c'est également à nos professeurs qu'il faut redonner envie de prendre le chemin de l'école, dans un contexte de crise aiguë des vocations, car l'école de la République n'existe pas sans ses hussards noirs. hussards noirs. Ces derniers ont besoin de confiance et de considération : pourtant, jamais les relations entre la communauté enseignante et son ministère n'auront été aussi dégradées et frappées du sceau de l'autorité et de la verticalité. Nous devons aussi leur fournir de bonnes conditions de travail : cela implique des créations de postes, mais aussi plus de formation continue, une meilleure protection et des moyens matériels.

Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, si nous ne réagissons pas, l'école publique, déjà mise à mal, sera bientôt devenue si fragile que notre système éducatif finira par ressembler dangereusement à celui des États-Unis : un système favorable aux plus aisés, bien loin de notre rêve républicain. Ne nous y trompons pas : si notre école publique et républicaine vacille aujourd'hui, ce n'est pas par manque d'autorité ou de flexibilité, mais bien parce qu'elle n'écoute pas assez les cris d'alerte de celles et de ceux qui la font vivre au quotidien ! La parole est à M. Cédric Vial. Madame la présidente,

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, Georges Bernanos avait eu ces mots désormais célèbres Hélas ! c'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents. » Madame la secrétaire d'État, il commence à faire froid ! Je voudrais ici évoquer notre politique de la jeunesse : celle que mène l'État, celle que se doit d'avoir notre nation. L'attention qu'une société porte à sa jeunesse est une attention portée à son avenir. La jeunesse n'est pas un état permanent ; ce n'est qu'une étape, un état provisoire dont tous sortent inégalement armés pour affronter la vie d'adulte et la vie en société. Notre politique de la jeunesse est donc non seulement un enjeu majeur pour cette dernière, mais aussi un enjeu national qui porte en lui les prochaines réussites ou les prochains échecs de notre modèle de société. La jeunesse ne dure pas, elle ne se recommence pas. Nous n'avons donc qu'une seule chance de réussir. Les jeunes consomment le présent ils sont l'avenir, mais ils ne le savent pas. C'est le rôle du politique que de donner du sens à cette période de la vie où l'on se prépare, où l'on se forme, où l'on apprend à devenir autonome, puis indépendant, où l'on apprend à être soi-même, mais aussi- ou « en même temps », si vous préférez, madame la secrétaire d'État -à faire partie d'un tout, d'une société organisée qui a déjà ses règles. Il y a alors deux manières d'envisager les choses que l'on pourrait formuler ainsi de quoi les jeunes ont-ils envie, ou besoin, et quelles réponses leur apporter ? D'autre part, qu'attend notre pays de sa jeunesse et de quelle politique en direction des jeunes a-t-il besoin ?

la mission budgétaire « Sport, jeunesse et vie associative » sont minuscules et ne concernent que quelques dispositifs ; ils ne sont pas même le petit bout de la lorgnette ! Une vraie politique de la jeunesse devrait évidemment porter sur l'éducation, la santé, la mobilité, la sécurité, l'emploi, la famille, l'innovation, le sport, le logement, ou encore la transmission des valeurs et des principes de la République. Mais pour chacun de ces enjeux, chaque ministre garde sa clé et personne- même pas vous, madame la Je veux ainsi dénoncer le manque coupable de vision interministérielle d'une vraie politique en direction de notre jeunesse. La somme de dispositifs n'a jamais fait une politique globale. globale. Certes, tout n'est pas noir au tableau ; il y a des points positifs, fort heureusement. Ainsi, les services civiques fonctionnent plutôt bien, même si une vision moins comptable et plus qualitative mériterait d'être mise en place, avec par exemple, pour chaque mission de service civique, une qualification ou une certification de compétences à la clé. Mais le Mais le SNU, le service national universel, est un cinglant échec de votre gouvernement. Il faudra le revoir de fond en comble ! Le dispositif « 1 jeune, 1 solution » fonctionne en revanche plutôt bien, mais le contrat d'engagement que le Gouvernement vient d'improviser avant les élections n'est qu'un variant du RSA jeune qui ne dit pas son nom la politique menée depuis cinq ans n'a pas permis de réduire les fractures qui existent, encore trop nombreuses chez nos jeunes. La lutte contre le décrochage scolaire est un point noir de votre bilan. Les actions de lutte contre la drogue, la délinquance juvénile et les violences, de manière plus générale, sont autant d'échecs. La perte de repères et de reconnaissance dans le projet et les principes républicains est encore plus flagrante. Plus de 52 % des jeunes et, en particulier, près de 78 % des jeunes musulmans ne reconnaissent plus l'intérêt de notre modèle laïque et remettent en cause, par exemple, le droit au blasphème. Nous avons le devoir de travailler à une politique qui permette à notre société de préparer son avenir, en n'oubliant personne au bord du chemin. Nous avons besoin de donner du sens à cette politique de la jeunesse pour que les intéressés s'y reconnaissent et comprennent les enjeux de notre nation tout entière. Nous avons besoin d'en discuter dans notre société et au Parlement.

À l'école, le dédoublement des classes de CP a plutôt bien réussi, mais cela ne suffit pas : il faudrait être capable de passer à une prise en compte encore plus individualisée des accompagnements éducatifs, pour ne pas laisser des difficultés se poursuivre de trimestre en trimestre et d'année scolaire en année scolaire. Là encore, la réponse passe par plus de déconcentration. Les réponses doivent pouvoir être adaptées par rectorat et plus probablement par département. Le système national de recrutement des enseignants impose aujourd'hui plus de contraintes qu'il ne résout de problèmes. Il faudrait être capable de concevoir des politiques de ressources humaines plus locales en développant, par exemple, les profils de poste à mission. mieux prendre en compte les évaluations des chefs d'établissement ou des cadres intermédiaires dans la politique d'affectation. Ainsi, on concentrera les efforts là où ils sont le plus attendus pour ne laisser, encore une fois, personne au bord du chemin. Madame la secrétaire d'État, la politique de la jeunesse dans notre pays est bien une politique en direction des jeunes, mais elle doit aussi être une politique pour la France : celle d'aujourd'hui et, surtout, celle de demain

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la crise de la covid-19 a changé beaucoup de choses ; elle a remis en question de très nombreuses certitudes et a mis en exergue certaines lignes de fracture dans notre pays. Nous avons évoqué à plusieurs reprises dans notre hémicycle les problématiques rencontrées par la jeunesse. Je salue la tenue de ce débat, qui permet une nouvelle fois d'aborder ces problématiques. Maintenant, nous espérons simplement que les actions suivront. Une étude menée par le réseau Animafac révèle que 35 % des jeunes considèrent que la crise sanitaire a affecté leurs aspirations futures ; 60 % d'entre eux estiment faire partie d'une « génération sacrifiée

Malgré de très bons résultats scolaires et une belle mention au baccalauréat, il n'a pas obtenu ses premiers voeux sur Parcoursup et se retrouve sur une liste d'attente. Ne pouvant aller étudier à l'étranger, pour des raisons financières, il se retrouve contraint de s'inscrire par défaut en licence, pour ne pas faire une année blanche.

Les fins de mois sont difficiles ; du fait de la crise sanitaire, il n'arrive pas à trouver de petit boulot. Il aurait bien eu besoin d'un ticket restaurant étudiant pour se nourrir le soir et le week-end, mais le Gouvernement ne souhaitait pas le mettre en place. Je suis désolé, madame la secrétaire Il se résigne à aller aux Restos du Coeur. Il n'en parle pas à ses parents, car il ne veut pas les inquiéter. Au plus fort de la crise de la covid-19, ses journées se résument à des cours en visioconférence, procédé qui en diminue largement l'intérêt. Les échanges avec les enseignants sont très limités. Il ne connaît pas encore ses camarades de promotion pas de soirées étudiantes, pas d'activités communes. Sa vie sociale est réduite à la portion congrue. Il se demande réellement s'il vaut la peine de continuer ses études. Un sentiment de découragement l'envahit, d'autant qu'il a lu des témoignages de jeunes diplômés de master 2 qui, après cinq ans d'études, ne trouvent pas d'emploi dans leur domaine

Malheureusement, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et la covid-19 ont changé la donne. Il y a beaucoup moins de places et il ne pourra peut-être pas partir. Notre étudiant se dit qu'il n'arrivera pas à accomplir ses objectifs de vie. Il remet beaucoup de choses en question. La souffrance de cet étudiant, madame la secrétaire d'État, est celle de milliers d'autres depuis le début de cette crise sanitaire

La parole est à Mme Béatrice Gosselin, pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, plus de 8 millions de Français ont entre 11 ans et 19 ans. Ce ne sont plus des enfants, pas tout à fait des adultes. Les temps de transition sont toujours des temps d'anxiété. En outre, d'après Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste, la précarisation croissante des liens sociaux, s'accompagne d'un état grandissant d'insécurité psychique. des dernières études sur le changement climatique, qui leur dessinent un avenir incertain, et la crise sanitaire, économique et sociale de ces deux dernières années angoissent particulièrement notre jeunesse. Mais une autre question inquiète aussi le jeune qui songe à l'adulte qu'il sera demain : quelle formation suivre pour s'insérer dans la vie active ?

Alors que 15,1 % des jeunes Français de 15 ans à 34 ans sont sans emploi, sans diplôme et sans formation, ce taux n'est que de 9,9 % de l'autre côté du Rhin. Le contrat d'engagement jeune a pour objectif de faire baisser le chômage, mais il convient de rappeler que ce dispositif tente de combler les défaillances de notre système scolaire, avec 95 000 jeunes qui sortent chaque année sans qualification. aussi que le premier versement de ce dispositif interviendra à six semaines du premier tour des élections présidentielles. Serait-ce un hasard ? Pour faire baisser radicalement le nombre de jeunes sans formation, il me paraîtrait plus efficace de privilégier l'apprentissage, comme dans le système allemand. Cet enseignement pratique, véritable facteur d'insertion et de mobilité sociale, connaît aujourd'hui des résultats réels. Mais il faut être beaucoup plus ambitieux. C'est assez paradoxal alors qu'il est une voie d'accès efficace à l'emploi durable et qu'il a permis en France la formation d'un chef d'entreprise sur deux, l'apprentissage, porté par l'artisanat, souffre toujours d'une mauvaise image. On l'assimile trop souvent, en effet, à un échec du système scolaire traditionnel. Face au chômage élevé et persistant des jeunes les moins diplômés, les gouvernements successifs ont tenté de mettre en place plusieurs mesures pour favoriser leur insertion sur le marché du travail. Malheureusement, le système actuel manque de lisibilité et certaines aides sont peu mobilisées.

appliquer la règle dite « des 3-6-9-12 » : pas de télévision avant 3 ans ; pas de console de jeux avant 6 ans, et avec un usage contrôlé ensuite ; pas d'internet sans être accompagné avant 9 ans ; et un accès internet seul, uniquement à partir de l'entrée au collège, vers 11 ans Une surexposition aux écrans peut entraîner des retards de langage, des troubles cognitifs, des troubles du comportement comme l'agressivité ou le repli sur soi, mais aussi des problèmes physiques : la vue et l'audition peuvent être altérées plus vite chez les enfants qui passent beaucoup de temps devant les écrans- entre 12 ans et 15 ans, un jeune sur dix souffre de baisse auditive. La musique trop forte, trop longtemps diffusée, entraîne des pertes d'audition irréversibles et la surdité, même partielle, est un facteur d'isolement supplémentaire. L'accès à internet apporte le meilleur- des connaissances, un réseau illimité d'informations -, comme le pire, car c'est aussi, malheureusement, le lieu du cyberharcèlement. Les jeunes, adeptes de ces relations virtuelles aux milliers d'« amis » se trouvent parfois victimes de harcèlements sexuels ou raciaux aux conséquences qui peuvent être dramatiques. Le numéro d'écoute 3018, qui permet de signaler des comportements délictueux, ne résout pas le déficit persistant de professionnels en pédopsychiatrie ou le manque d'accueil dédié, notamment en zone rurale. Il est dommage que le cyberharcèlement ne soit pas une infraction réprimée en tant que telle par la loi française. La situation actuelle doit nous inciter à apporter des réponses d'urgence face à cette crise vécue par notre jeunesse. C'est le seul moyen, j'en suis convaincue, de prévenir l'apparition d'une génération sacrifiée. La parole est à Mme la

Hélas, les objectifs fixés en termes d'effectifs pour 2021 ne devraient pas être atteints d'ici à la fin de l'année. En effet, il y a peu, pour le mentorat, seuls 45 000 jeunes étaient inscrits sur les 100 000 envisagés. national universel, le même constat peut être observé avec moitié moins de recrues que prévu. Dans ces conditions, bien évidemment liées à la pandémie, et en période préélectorale, est-il prudent de promettre, comme c'est le cas dans le projet de loi de finances pour 2022, des cibles d'effectifs trop ambitieuses ? En outre, ne faudrait-il pas évaluer ces dispositifs avant de les généraliser quoi qu'il en coûte ? Un peu de modestie budgétaire à leur égard aurait permis de soutenir d'autres secteurs également fragilisés par la crise sanitaire. Je pense aux colonies de vacances et, plus largement, à l'accueil des plus jeunes pour lesquels la formation des animateurs et encadrants a pris un sérieux retard, ce qui entraîne d'importantes difficultés de recrutement. Or le prochain budget entérine une baisse de 18 % des crédits consacrés aux examens et certifications, là où il aurait fallu les stabiliser

Outre qu'il interfère avec les choix politiques des élus, il durcit les conditions de contractualisation et hypothèque certains financements. Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous rassurer les élus locaux sur la préservation de leurs politiques contractuelles en direction de l'enfance et de la jeunesse ?

trop lourdes sur les victimes. Le cyberharcèlement aggrave encore le phénomène, car il abolit les frontières de l'établissement pour ne laisser aucun répit aux enfants harcelés. Et les réseaux sociaux agissent peu dans la lutte contre les actes de malveillance sur internet. Il faut que la présidence française de l'Union européenne porte ce dossier au niveau européen et que, parallèlement, ce juste combat soit déclaré grande cause nationale 2022-2023. Le harcèlement scolaire est l'affaire de tous, et à ce titre l'intervention du Président de la République du 18 novembre dernier a au moins permis d'aborder la question, même si les mesures annoncées sont bien insuffisantes. II n'y a pas de remède miracle pour lutter contre ce fléau, et il ne doit pas y avoir de fausse polémique entre nous puisque, depuis plus de dix ans, tous les gouvernements se sont mobilisés sur cet enjeu. Cependant, je regrette que ni le Président de la République ni le ministre Blanquer n'aient évoqué les travaux du Sénat sur la question, et particulièrement le rapport de la mission d'information que j'ai eu l'honneur de présider aux côtés de notre collègue rapporteure Colette Mélot. Pas un mot sur la nécessité de plus de personnels médico-sociaux dans les établissements ; pas un mot non plus sur la nécessité d'une formation accrue des personnels des établissements pour faciliter la détection des signaux faibles pas un mot, enfin, sur les mesures simples de communication à destination des élèves. Ces quelques mesures sont extraites des trente-cinq propositions unanimes de la mission d'information sénatoriale, qui sont le fruit d'un constat : les dispositifs existent,

Quand allez-vous enfin vous emparer des propositions de notre mission, propositions qui sont à la fois concrètes, réalistes et applicables immédiatement, pour peu que la volonté politique soit là ? La parole

Les valeurs intangibles, le sens du collectif, l'esprit civique qui y sont inculqués forment la clé de voûte indispensable à la cohésion de notre société. L'un des piliers de cet apprentissage est l'éducation morale et civique, une matière à part entière depuis la réforme de 2015. Cette matière mériterait encore des ajustements, me semble-t-il. Il conviendrait d'abord d'augmenter le nombre d'heures qui y sont consacrées ou, à défaut, de prioriser son contenu au regard de l'ampleur du programme. Par ailleurs, je pense souhaitable de renforcer le programme « Apprendre ensemble et vivre ensemble » à l'école maternelle, en insistant notamment sur la prévention et la lutte contre le harcèlement scolaire, qui touche aussi les très jeunes enfants. Le ministre de l'éducation nationale a annoncé l'année dernière vouloir valoriser l'engagement des élèves dans le cadre d'une réforme du brevet des collèges. Cette idée me semble très intéressante : est-elle toujours d'actualité ? Le cas échéant, sous quelle forme l'envisagez-vous ? Je pense qu'il faudrait également valoriser l'engagement des citoyens, notamment le bénévolat des élèves de lycée au travers de Parcoursup, en prévoyant une rubrique dédiée dont les algorithmes pourraient tenir Enfin, je souhaite attirer votre attention sur l'importance de développer le mentorat entre lycéens et jeunes diplômés des grandes écoles, pour contrer l'éloignement social et géographique des élèves des écoles les plus sélectives de notre pays, souvent parisiennes. En milieu rural, nous constatons une forte autocensure chez des élèves pourtant prometteurs. Institutionnaliser le mentorat serait un moyen de lever cet obstacle, tout en favorisant la réussite de tous les élèves. Nous sommes là au coeur de l'idéal républicain et de la promesse républicaine.

qui pose la question du brevet, du service national universel et de la reconnaissance des engagements bénévoles dans Parcoursup. Aujourd'hui, il existe une première rubrique, mais sincèrement nous pouvons aller beaucoup plus loin en termes de reconnaissance du bénévolat et de l'engagement, que ce soit dans le cadre de la démocratie scolaire-

la réforme du baccalauréat n'est pas encore arrivée à son terme qu'elle engendre déjà deux difficultés d'importance : sur le parcours des élèves et leur orientation, ainsi que sur les conditions de leur évaluation. Point de départ de la réforme, l'organisation par spécialités pouvait permettre de décloisonner le cursus des élèves pour en finir avec la rigidité des anciennes filières. Malheureusement, vous le savez, l'offre de spécialités varie considérablement d'un établissement à l'autre. Pire, le retour des options crée de nouveaux besoins financiers qui vont encore aggraver la baisse du nombre de spécialités enseignées dans les lycées. Cette situation entraîne une véritable inégalité des chances entre les lycéens, dont nombre ne pourront suivre le cursus de leur choix. Moins cohérent ou moins complet, le profil de ces bacheliers fragilisera leurs candidatures auprès des établissements de l'enseignement supérieur. Concernant le contrôle continu, sa forme actuelle présente deux inconvénients. Il confère une dimension locale au baccalauréat, qui devait pourtant demeurer un diplôme national. Chacun connaît les fortes disparités de niveaux persistant d'un établissement à l'autre et sait qu'elles engendrent des barèmes de notes différents. Cela introduit un nouveau biais dans le dossier des élèves, avec des conséquences certaines sur leur traitement par Parcoursup. De plus, le contrôle continu nourrit les pressions que subissent un nombre croissant de professeurs, à qui des parents d'élèves, certes anxieux, mais parfois vindicatifs, reprochent leur notation.

mon collègue Thomas Dossus a abordé le sujet de la précarité grandissante des jeunes et de l'avenir que nous leur offrons. Cet avenir est étroitement lié à celui des étudiants et des universités françaises. J'aimerais vous donner deux chiffres marquants. Entre 2017 et 2022, le budget de l'enseignement supérieur rapporté au nombre d'étudiants a baissé de 7 % et le taux d'encadrement a, lui, chuté de 15 % en dix ans. Nous savons que l'enseignement supérieur fait face à une augmentation importante du nombre d'étudiants. Elle est due en grande partie au boom démographique. L'évolution des effectifs, et donc des besoins, aurait dû être anticipée. Il est toujours possible de changer de vision et de réagir afin d'offrir de réelles perspectives à notre jeunesse. Le Gouvernement ne peut plus ignorer le manque de budget des universités. Les présidents d'université nous le disent : ils sont dans une situation financière préoccupante et n'ont plus aucune marge de manoeuvre budgétaire, pourtant nécessaire pour l'accueil de nouveaux étudiants. Le nombre de places, notamment à l'entrée en master, n'a pas suffisamment augmenté et beaucoup d'étudiants se retrouvent sans solution de poursuite d'études. Bien d'autres n'accèdent pas à la filière qu'ils souhaitent et subissent une orientation par défaut. La nouvelle sélection en master risque d'aggraver les inégalités et de contraindre encore davantage les choix des étudiants. Quand le Gouvernement proposera-t-il un budget décent pour l'enseignement supérieur français afin de donner la possibilité à tous les jeunes qui le souhaitent de poursuivre les études de leur choix ? La parole

L'accompagnement pédagogique et psychologique participe aussi de la réussite des étudiants : plus de 10 000 étudiants ont bénéficié d'aides gratuites de psychologues depuis mars 2021.

Madame la secrétaire d'État, la semaine dernière, l'académie de Lille annonçait la fermeture de 667 classes, dont 511 dans le seul département du Nord, soit près du double par rapport à la semaine précédente. Le Nord et le Pas-de-Calais étaient les deux départements les plus touchés après l'académie de Versailles. Contrairement à ce que vous avez défendu pendant des mois, malgré toutes les études scientifiques et les retours de terrain, l'école est donc bien un haut lieu de contamination pour les enseignants, les personnels, les enfants, et donc les familles. Au vu de la situation, je dois admettre que je partage l'inquiétude et l'incompréhension des organisations syndicales face au protocole sanitaire que Jean-Michel Blanquer a annoncé la semaine dernière. Ainsi, dans le but de limiter les fermetures de classe, un cas positif ne vaudra plus fermeture de celle-ci. Seuls les enfants ne pouvant pas fournir un test négatif seront placés à l'isolement. Bien évidemment, il n'est jamais bon pédagogiquement de fermer des classes durant une semaine prend le risque que les enfants accumulent du retard. Mais nous ne pouvons que nous interroger sur le bien-fondé d'un allégement du protocole sanitaire au moment même où l'épidémie accélère, au risque d'exposer un peu plus les enfants et le corps enseignant à la maladie. ce protocole est flou et donne le sentiment de laisser les enseignants, les parents, les directions d'établissement livrés à eux-mêmes face à l'épidémie. Au fond, madame la secrétaire d'État, comme beaucoup, nous nous interrogeons sur la finalité de ce nouveau protocole : son objectif ne serait-il pas de garder les parents au travail et de faire baisser les chiffres ? Or il faut rappeler que nous parlons de la santé d'enfants non vaccinés, et dont le taux d'incidence est 1,8 fois supérieur à l'ensemble de la population.

Face à ce constat, de nouveaux dispositifs comme le mentorat ou le renforcement de la formation de tous les professeurs à l'orientation ont été mis en place. Néanmoins, la catastrophe éducative qui touche notre pays persiste, et les inégalités sociales se reproduisent dans le parcours scolaire. Ainsi, en 2018, 93 % des élèves ayant une mère diplômée de l'enseignement supérieur obtiennent le baccalauréat, contre 58 % de ceux dont la mère est sans diplôme. De même, 67 % des enfants de cadres obtiennent un diplôme de l'enseignement supérieur au-delà de la licence, contre seulement 16 % des enfants d'ouvriers.

Parmi ces recommandations, certaines nous semblent indispensables : accélérer le dédoublement des classes de grande section en éducation prioritaire et étendre le dédoublement des classes jusqu'au CE1 au-delà des QPV ; améliorer la formation des enseignants afin de favoriser une meilleure prise en compte des élèves les plus en difficulté ; étendre le dispositif Devoirs faits dans les écoles élémentaires et l'adapter aux contraintes des transports en commun dans les territoires ruraux. Madame la secrétaire